La séance est reprise bonjour chers collègues, bonjour monsieur le Ministre, l'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances dans les discussions des articles que nous sommes parvenus à l'article. Nous allons examiner l'article d'équilibre et l'État a sur les voies et les moyens, mais Monsieur le Ministre, vous venez de déposer un amendement que la commission est en train d'étudier donc je vous propose de suspendre la séance avant que vous ayez un mot à dire. Oh merci madame la présidente, effectivement on arrive à l'issue de cette partie, hein, on doit examiner l'adaptation à la fois de l'article liminaire et de l'article, l'équilibre, l'article d'équilibre, c'est en quelque sorte la facture de la discussion qu'on a eu dans la première partie et on doit intégrer dans l'équilibre et dans les chiffres, tous les amendements qui ont été adoptés, qui ont évidemment un impact sur le sol de public sur la dépense publique sur la dépense fiscale il y a une grande masse d'amendements qui ont été adoptées, y compris encore ce matin, ce qui veut dire que les services de Bercy qui ont travaillé pendant toute l'heure du déjeuner pour actualiser l'article d'équilibre et je veux vraiment leur rendre hommage, ils ont travaillé tout le déjeuner pour intégrer les amendements qui ont été adoptés, encore ce matin aux données chiffrées, que l'on doit présenter dans certains article d'équilibre, ils l'ont envoyé seulement il y a quelques minutes à la commission, ce qui explique l'absence je crois du président et du rapporteur général qui sont encore en train de l'examiner, donc je suis vraiment auprès de chacune et chacun d'entre vous pour ce délai mais il faut que l'article d'équilibre soit le plus proche possible du chiffrage des amendements qui ont été adoptées par cette assemblée, si on ne faisait pas ça voudrait dire qu'on ne respecte pas les votes qui ont eu lieu et qu'on intègre pas dans la comptabilité, les différents amendements qui ont été adoptés, donc j'imagine madame la présidente, qu'il va falloir suspendre un peu avant. C'est ce que j'ai annoncé, Monsieur le Ministre, donc je vais suspendre la séance pour dix minutes minimum dix minutes, un quart d'heure, hein, voilà c'est je, je vous rappellerai, peut-être un peu plus tôt, écoutez bien les les sonneries en tout cas ne vous éloignez pas trop, mais voilà, on attend la fin de la la commission des finances à tout à l'heure, cher collègue, Monsieur le Ministre, merci.

à nouveau jusqu'à 17 heures. Donc, nous nous donnons rendez-vous à 17 heures dans une heure, pour reprendre la séance tout à l'heure, chère collègue, la séance est suspendue.

Cher collègue, Monsieur le Ministre, la séance est reprise, je donne la parole immédiatement au président de la commission.

pour permettre d'abord de d'avoir une une bonne lecture de l'article d'équilibre qui a été proposé à 14 heures 30, 14 heures 45, même je crois par par le gouvernement et le temps évidemment, pour le rapporteur général de faire son travail d'analyse

et deuxième 2ème point vous dire qu'avec un peu de réussite, et avec un peu de maîtrise du débat, nous serions susceptibles de pouvoir démarrer une première mission à dix-huit heures trente mais c'est leur ultime pour pouvoir démarrer la première mission et donc j'engagerai, comme d'habitude, tout le monde, air à regarder pour maîtriser ce temps voilà, merci beaucoup, madame la présidente. nous avons un amendement 581 présenté par Monsieur Breuiller. Merci madame la présidente, c'est un amendement très intéressant qui vise à améliorer notre capacité à analyser les enjeux de la crise écologique et leur prise en compte dans le budget, mais je le retire parce que je pense qu'après la longue interruption de séance, qu'il y a eu les conditions du débat sur cet amendement ne seront pas les meilleurs.

Merci madame la présidente, c'est donc un amendement classique dans un PLF qui vise à l'issue de l'examen du texte de proposer l'article d'équilibre qui tient compte de l'ensemble des décisions décisions que cette assemblée a prise dans le courant de l'examen des amendements qui ont été votées sur la première partie sur la partie donc recette de ce PLF je ne vais pas revenir dans l'intégralité du détail de ce qui a été votée, on a eu plus d'une semaine de débats, on peut dire que dans les mouvements significatifs : il y a eu le choix de ne pas supprimer la CVAE et donc de revenir sur la suppression proposée de la CVAE au bénéfice des entreprises et notamment de l'industrie et donc c'était quatre milliards de recettes qui devaient que nous devions perdre entre guillemets l'an prochain, qui finalement, dont la dégradation n'est pas intégré dans le sol, on va dire que c'est un plus 4 milliards de recettes par rapport à la copie initiale du gouvernement, ensuite il y a un certain nombre d'amendements de de recettes qui ont été adoptés notamment la suppression enfin le le relèvement du barème pour les droits de succession, 3 milliards d'euros, un certain nombre d'amendements sur des baisses de TVA que je globalisera autour de 700 millions d'euros avec la baisse de TVA à 5 5 sur la margarine 115 millions d'euros avec la baisse de la TVA à 5 5 sur la filière équine qui est chiffré à 190 millions d'euros, la baisse de la TVA sur les transports de voyageurs, 350 millions d'euros tout ça faisant un paquet TVA qui coûte aux finances publiques 700 millions d'euros il y a ensuite, décision qui a été prise avec un amendement sur le si je résume le relèvement du crédit d'impôt pour la garde d'enfant 250 millions d'euros. Le relèvement du plafond de liesse PME 320 millions d'euros, tout ceci faisant que et pardon un sous-amendement un sous-amendement qui a été porté par adopter qui était défendu par Madame Lavarde, il faut se souvenir quand on a débattu de l'amendement du gouvernement pour élargir la crie la contribution sur la route en fermant infra-marginale des énergéticiens, vous savez que j'ai défendu un amendement du gouvernement pour que nous puissions capter davantage de superprofits des énergéticiens et passé le rendement de ce mécanisme européen de 7 milliards à 11 milliards d'euros, c'est un amendement, je le concède, qui est arrivé tardivement, que c'est un mécanisme récent qui a été trouvé au niveau européen et que, forcément, on se souvient Monsieur Savoldelli des conditions dans lesquelles ça s'est fait il y a un certain nombre, un certain nombre de sous-amendements ont été déposés à cet amendement du gouvernement, ils ont été débattus discuter ces sous-amendements étant arrivés très tardivement, je n'ai pas pu vous avez pas posé la question, par ailleurs, mais je n'ai pas pu, au moment où j'ai répondu et donner mon avis sur les sous-amendements vous communiquer le coût de ces sous-amendements, il se trouve qu'un des sous-amendements qui étaient proposés par le groupe Les Républicains auquel le rapporteur général et moi-même avons avions donné un avis défavorable, a été adoptée, on s'est rendu compte hier soir quand le chiffrage a été fait que ce sous nos amendements coûtait 6 milliards d'euros, ce qui en fait des sous-amendements les plus cher je pense de l'histoire du PLF, ce qui fait qu'il y a une dégradation très forte du solde, à l'issue de l'examen, et que le solde public arrive au lieu des 5 % qui avait été présenté dans le cadre du PLF initial à 5,2 pour 100 de déficit l'an prochain, voilà l'article d'équilibre telle qui vous est proposé, telle qu'il est immédiatement issue pour le coup c'est statistiques c'est mathématique des votes qui ont eu lieu dans cette assemblée. Merci, monsieur le rapporteur, votre avis s'il vous plaît. Alors Monsieur le ministre, on va en prendre, enfin, j'ai proposé qu'on en prenne acte et je rendrai donc un avis de sagesse, mais je vais préciser tout de suite parce que je vais proposer des amendements. Je je vais revenir effectivement sur à la fois le le le déroulement de nos travaux et ce ce qu'a précisé encore le le président en ouverture de cette séance. On a quand même dans ce dans ce débat budgétaire du PLF, dont je rappelle qu'il a été déposé, elle présente en Conseil des ministres le 26 septembre de cette année, on a quand même des difficultés encore à cette heure pour avoir sur des articles de ce projet de loi de finances pour 2023 des estimations précises. Donc on va pas se renvoyer la balle, c'est pas le c'est pas le ça n'est pas l'objet, seul, mais je le signale, quand même, parce que ça nuit à la qualité de nos travaux. Vous dans les amendes, les, comment dirais-je, la 2ème délibération que je vais proposer, je le dis tout de suite au nom de la commission, il y aura donc une demande de 2ème délibération sur 3 articles, le 3 octobre des siestes eux le 3 nouveaux des et le 4 du haut des sieste et évidemment l'article liminaire L article d'équilibre pour pouvoir tirer les conséquences de cette seconde délibération et c'est effectivement vous qui le déposerai mais Monsieur le Ministre, pour au moins 2 de ces 3 articles, nous n'avons pas eu de communication et tant et si bien, vous l'avez dit, par exemple sur la le sous-amendement qui est estimé depuis hier soir, vous l'avez dit vous-même, à 6 milliards finalement, on a une vraie difficulté, vos services il y a 15 jours, 3 semaines, un 1er document sur ce sujet de plus de 30 pages. Puis une bonne dizaine de jours à près de 30 pages, le document est passé à 15, donc il fallait, il a fallu retravailler et vous l'avez dit, y compris dans le débat, tout n'est pas encore stabilisé, raison pour laquelle, d'ailleurs j'avais demandé l'avis du gouvernement, raison pour la quelle vous venez de dire que vous n'aviez pas répondu ou pas pu répondre mais peu importe, c'est pas, c'est pas un jugement, ça n'est pas un reproche sur ce sujet, convenez que de faire confiance au ministre et donc au gouvernement pour pouvoir travailler et ne pas bloquer la machine, finalement, il y a, on a un espèce d'effet boomerang qui revient, qui nous revient, ça a un côté désagréable mais je pense que c'est désagréable pour tout le monde parce que ça pose une difficulté, c'est de pouvoir prendre une décision. une envie de confiance mais sans avoir les chiffres parce que sinon on bloque, et vous voyez que si on avait bloqué la probabilité c'était ça aurait été dire ils font un refus d'obstacle, ils veulent pas, ils font de l'obstruction, ça n'est pas l'esprit de notre assemblée, et là, je pense, par le dire, toutes tendances confondues, vous l'avez vu hier encore sur des sujets importants, notamment sur le filet de sécurité, faut, il faut convenir que c'est ça, c'est difficile de pouvoir bien travailler et quelque part bien légiférer dans ces conditions, voilà je, je, vraiment, je tenais à le dire, cette une difficulté à laquelle quand même, il faudra pouvoir à l'avenir répondre parce que moi je vous le dis, en tous les cas dans dans l'exercice de la fonction si ça venait à se reproduire, nous prendrions à ce moment-là, des précautions et puisqu'on en est là, Monsieur le Ministre, je veux vous dire que qu'avec le présent Claude Raynal, dès maintenant, je vous annonce qu'au nom de la commission des finances notamment, mais je pense de notre assemblée, nous vous proposerons et nous vous demandons de bien vouloir intégrer le fait que sur l'amortisseur électricité dont on a toujours pas non plus connaissance cet amortisseur électricité qui va, comment dirais-je, produire des effets pour les collectivités, mais aussi pour nos entreprises, hé bien, comme on n'a pas les éléments on on demande à être associée le plus tôt possible et on procédera chaque trimestre à des contrôles sur pièces et sur place, parce que mon intuition me fait craindre des vraies difficultés, ça n'est pas un une c'est une précaution que nous voulons prendre, nous voulons qu'en tous les cas, notre assemblée, le Sénat et le maximum d'éléments pour nous permettre, s'il devait y avoir un moment des difficultés pour des raisons que vous ignorez, et moi aussi et je souhaite pas qu'il y ait des difficultés et que nous puissions avoir le meilleur niveau d'information possible parce que on sent comment dirais-je le le sujet prendre une, comment dirais-je, une certaine ampleur dans des inquiétudes de nos populations, or nous devons-nous être finalement des des modérateurs, on est là pour faire le lien avec les élus, les entreprises et nos concitoyens, donc on vous propose d'ores et déjà sur ce sujet, plus particulièrement, et notamment de l'amortisseur de prendre acte et j'espère que vous comprenez bien que l'essence de notre démarche.

ah, vous n'avez pas parlé sur l'amendement en seconde lecture et que le il y aurait ensuite les conséquences se retirer à l'issue. Je sais, c'est moi, hein, j'avait pas de souci, j'ai juste lu la la feuille d'après-midi, donc on en est à l'amendement.

Tout avant et explications de vote sur l'amendement moi je, je m'associe effectivement remarque du rapporteur général je, je, j'avoue que j'ai beaucoup de mal et on a beaucoup de mal à suivre malheureusement avec les informations dont on dispose, monsieur le Ministre, c'est pas que vous, hein, je dirais que nous, depuis quelques années, de, de, de sénateurs on, on constate qu'on a beaucoup de mal à avoir les informations et avoir le détail des informations alors moi j'avais déposé un amendement qui a été adoptée sur les plus-values immobilières, vous m'aviez annoncé que ça coûtait 4 milliards je recherche dans les dans les chips, je ne les vois pas ces 4 milliards, je les avais contestée et je pense que ça ne coûte pour moi rien en tout cas sur les estimations que j'avais fait un peu sommaire, mais j'avoue que c'est compliqué de de bien légiférer quand on a aussi peu d'informations et sur sur la taxation infra-marginal des des électriciens, moi j'ai on on a compris qu'il y avait aussi beaucoup de sociétés qui en fait dénoncer les contrats, on on ne sait pas jusqu'où ça va aller, parce que s'il y en a quelques-unes qui le font, pourquoi elle ne ferait pas toutes parce qu'on a quand même pas mal de produits qui sont liées à ces contrats, il y a 17 milliards ou 19 milliards je sais plus cette année qui sont liés, normalement, a assez au fait que l'électricité étant à un niveau très élevé, on a des recettes supplémentaires mais si toutes les sociétés contrat on a plus de recettes et finalement, on avait l'impression qu'on avait substitué la taxation infra-marginal aux recettes qu'on perdait mais honnêtement, on reconnaît pas du tout là, moi je vois 6 milliards je sais plus ce qu'il y a de l'autre côté, donc c'est vrai que moi, je ne vois pas personnellement, comment je peux voter cet article d'équilibre, compte tenu de ces informations-là quoi oui je, je suis dans le flou artistique et ça me paraît très compliqué, alors je comprends la vie de sagesse du rapporteur, mais pour moi en tout cas c'est j'ai j'ai du mal à me déterminer par rapport à cet article d'équilibre. Merci monsieur le président, la parole est à monsieur kaput pour explication de vote. Clair. Oui, madame la présidente, très rapidement, ce que je veux pas allonger les débats, on est tous un peu fatigué et puis on a tous travaillé dans des conditions effectivement d'urgence particulière, je ne vois pas dans l'amendement de 2 mention du coût lié à l'amendement de la commission sur sur l'élargissement du filet de sécurité or manifestement ça a nécessairement un coût qui est relativement important, en tous les cas, c'est ce que le gouvernement nous a dit, pour ah la pour rejeter les les amendements qu'on avait déposé et et la et et donner un avis négatif sur l'amendement de de du rapporteur général donc ça me surprend qu'il y ait pas de référence pas de référence à ce surcoût dans dans l'amendement du gouvernement. Merci madame présidente, je vais essayer de répondre sur la méthode, on arrive à la discussion sur le PLF en séance, il y a 1700 je crois amendements qui sont déposés à partir de là, les services de Bercy évidemment ce qu'il cherche à faire c'est chiffré le plus possible les amendements pour que moi, en tant que ministre au banc je puisse informer le Parlement, le Sénat sur le coup de chacun des amendements, vous imaginez bien que 1700 amendements à chiffrer en quelques jours, ça demande un travail colossal, comment on procède : on prend les amendements pour lesquels on voit que la Commission va donner un avis favorable, donc on se dit qu'ils ont, a priori, beaucoup de chance d'être adoptée au Sénat, on part de ça pour les chiffrer ça n'empêche pas qu'il y a quand même des amendements pour lesquels on n'a pas l'intégralité du chiffrage quand on arrive dans l'hémicycle on cherche au maximum à pouvoir chiffrer mais mais tous les amendements ne peuvent pas être être chiffrées immédiatement au moment de la discussion, vous m'avez interrogé Monsieur de La Haye sur le chiffrage de votre amendement sur les plus-values et pourquoi est-ce qu'il n'a, il n'est pas dans l'article d'équilibre, la raison pour laquelle il n'est pas dans l'article d'équilibre, c'est qu'il n'a pas un impact en 2023 mais en 2024 du fait des modalités d'entrée en vigueur de votre amendement pour autant le chiffrage, j'avais parlé de Big bang du marché de l'immobilier, vous imaginez que ça nécessite un chiffrage très poussée, très nourris, j'ai de premières informations sur le chiffrage que je peux vous communiquer, si vous le si vous le souhaitez, pour vous donner quelques ordres de grandeur, de son impact financier et pour que le Sénat puisse apprécier donc l'impact du vote, la seule baisse des taux d'impôt sur le revenu, représente un coût de l'Ordre de 600 millions d'euros, la baisse des prélèvements sociaux pourrait représenter une perte d'un milliard d'euros pour la sécurité sociale, on est un milliard 6 la suppression de la taxe sur les plus-values exceptionnelles ajouterai un coût additionnel de 100 millions d'euros, donc un milliard enfin l'amendement propose de remplacer les abattements pour durée détention par un coefficient d'érosion monétaire le chiffrage de cette mesure est complexe, car il dépend notamment de l'inflation, plus l'inflation est élevé, plus la mesure et coûteuse, évidemment, faits c'est il faut vraiment se projeter sur les niveaux d'inflation prévue en 2024 ce qui est aujourd'hui assez hypothétique, mais pour vous donner un ordre de grandeur des estimations réalisées en 2019 nous avait amené à conclure avec une inflation stable à 2 beaucoup moins élevé que ce que nous connaissons aujourd'hui la mesure coûtait déjà 700 millions d'euros, donc on serait à 2 milliards 400 millions d'euros il y a encore des dimensions qui reste à chiffrer, mais ça n'a pas d'impact sur 2023 puisque la mesure entrerait en vigueur en 2000 24 sur la cri je vous confirme que dans le mécanisme qu'on a aujourd'hui de CSPE qui nous permet de récupérer la rente infra-marginal des énergéticiens du renouvelable, on chiffre à 4 milliards d'euros le coût des énergéticiens qui ont unilatéralement quitter leur contrat pour ne pas avoir à rendre à l'État ce qu'ils doivent à l'État, du fait des contrats, mais que l'intégralité d'entre eux seront rattrapés par la nouvelle cri d'où une partie de l'élargissement des recettes prévues dans le cadre de la crise, donc à la fin il y a très peu de pertes pour l'État puisque ceux qui sortent du mécanisme CSPE on les rattrape, avec la contribution fera marginal européenne le la, la, l'amendement filet sécurité ne dégrade pas le déficit, parce que le solde public et calculé toutes administrations publiques, donc on vous avez un transfert de l'État aux collectivités locales, comme le déficit, le solde est calculé toutes administrations publiques, État, collectivités locales, Sécurité sociale, ça n'a pas d'impact facialement sur le solde public voilà pour les réponses que je pouvais apporter je précise quand même que cet amendement du gouvernement, raison pour laquelle le rapporteur général, a parlé d'en prendre acte, ne fait que mathématiquement, tenir compte de ce qui a été votée. On peut revenir sur ce qui a été votée, je crois qu'ensuite il y aura des seconde délibération présentera alors un nouvelle. Article d'équilibre, mais ça ne fait que tenir compte de ce qui a été votée et donc, et je précise que c'est très important qu'on ait un article d'équilibre cohérent avec les mesures qui ont été votées, parce que sinon il s'un risque constitutionnel sur le PLF. C'est arrivé une fois, je crois, dans l'histoire de la Ve République un PLF soit et après le PLF est pris par ordonnance, j'imagine que c'est pas le souhait des sénateurs et des sénatrices, donc c'est important que évidemment l'article d'équilibre soit cohérent avec le reste du texte. Merci, Monsieur le Ministre Monsieur là midi pour explication de vote.

extrêmement compliqué, il faut le dire, je le partage, nous le partageons tous ces tous parce que c'est ça représente un travail considérable, tant des services de la haute assemblée que des services du ministère des ministères concernés et moi je voudrais simplement et puis aussi des ça change tous les jours et les chiffres changent le solde budgétaire de l'État, au départ, il est estimé à son sang à moins 158 milliards d'euros, là, il passerait à sont moins de 162 milliards d'euros puis également à noter, puisque bon, il y a eu beaucoup de d'interventions liées aux collectivités territoriales c'est aussi une une majoration du prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales qui s'élèverait à plus 1 virgule 45 milliards d'euros, bon qui font suite aux amendements qui ont été je dirais adopté donc ce que je suivrai néanmoins toute tout à fait l'avis de la commission merci. Merci, je vais donc mettre aux voix avec hein, la vie de sagesse de la commission, l'amendement du gouvernement qui vote pour.

Il être adopté. Je vais mettre aux voix l'article d'équilibre, ainsi que l'État a annexé modifié par l'amendement que vous devenez de voter qui votent. Pour contre même vote, j'imagine que c'est le même vote même vote, il est donc. Ben si vous levez ni contre ni pour je pense que, à moins que vous vouliez, ne pas participer au vote, alors je demande : qui vote à ah Soyons formaliste qui vote pour. Il y a encore plus, qui vote contre. Qui s'abstient. Qui ne participent pas au vote. J'avais donc bien raison, vous êtes abstenue n'y a aucune non participation au vote parfait. Nous l'avons fait dans le formalisme requis en application de l'article 47 bis alinéa 1 du règlement, la commission demande qu'il soit procédé à une seconde délibération comme vous l'indiqué le rapporteur général des articles 3 Octo des sièges E 3 nouveau des siestes ah et Cadiot vif Yes et par voie de conséquence. Je pense que certains voudraient entendre ce que je dis donc si. Qui on peut parler un peu moins fort merci et par voie de conséquence de l'article liminaire et de l'article d'équilibre, cette seconde délibération et de droit, conformément à l'article 43 alinéa 5 du règlement lorsqu'il y a lieu à seconde délibération les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission qui doit présenter un nouveau rapport, la commission souhaite-t-elle une suspension de séance. Très bien les amendements adoptés par la commission ont été distribués ou en cours de distribution. Nous allons donc procéder. à la seconde délibération. Je rappelle au Sénat, les termes de l'article 43 alinéa 6 du règlement dans sa seconde délibération le Sénat statut seulement sur les nouvelles propositions du gouvernement ou de la Commission, présentée sous forme d'amendement et sur les sous-amendements s'appliquant à ces amendements,

celui qui résulte de l'adoption de l'amendement 309 de notre collègue Michel Calvez en fait cet article conduit à supprimer totalement le régime fiscal de l'assurance-vie, cet article additionnel pardon et non en fait, comme il était souhaité par son auteur, la seule dépense fiscale attachés aux produits d'assurance-vie de plus de 8 ans

Monsieur le ministre. 300 millions d'euros, c'était un relèvement de fiscalité sur l'assurance-vie, d'un milliard trois j'avais donné un avis défavorable dans ces conditions, je suis favorable à cette seconde délibération pour revenir dessus. Merci, monsieur le rapporteur, je mets donc aux voix cet amendement de suppression présentés par la Commission, qui vote pour. Qui vote contre. Qui s'abstient donc. Mais. Qui ne participent pas au vote. Très bien. L'amendement et donc adopté, monsieur le rapporteur général. De ce côté. Adopté dans sa suppression, bien sûr, l'amendement numéro 3. Donc, cet amendement vise à supprimer cette fois à l'article 3 nouveaux des sièges à du PLF qui était issu de l'adoption de l'amendement 12 quarante-quatre de notre collègue André Reichardt, c'est un article additionnel dont les conséquences se conduisent à rehausser de 50 % le montant des abattements en ligne directe pour l'application des dès MTG et de réduire le délai de reprise fiscale entre 2 donations l'estimation du coût pour les finances publiques environ 2 milliards d'euros. Merci, oui, c'est une seconde délibération qui revient sur l'amendement qui était porté par le groupe LR est je crois le sénateur Richard sur le relèvement de l'abattement des droits de succession, je précise simplement j'avais donné un avis défavorable à cet amendement, non pas sur le fond, parce que le président de la République s'est engagé dans le courant du quinquennat à relever le plafond de l'abattement sur les droits de succession, simplement le choix que nous avons fait pour l'année prochaine c'est de concentrer la baisse d'impôts sur la production des entreprises avec la CVAE donc je redis que l'engagement du président de la République sera tenu, mais nous sommes pas favorables à ce qu'il soit tenu dès 2023, raison pour laquelle je donne, je donne un avis favorable à cet amendement de suppression de cette mesure sur les droits de succession. Merci, je considère que c'est le même vote que le précédent. Je vais faire voter qui votent pour. Qui vote contre qui s'abstient qui ne participent pas au vote, parfait, c'était donc le même vote.

le sous-amendement 1727 de notre collègue Christine Lavarde qui tendent à traiter différemment les producteurs qui n'ont jamais le MLC de soutien public en ce qui concerne donc les, les, les, les, leurs dispositifs énergétiques demain notamment avec énergie renouvelable et qui présenterait un coût pour les finances publiques, cet amendement d'environ 6 milliards d'euros, je précise que la commission des finances qu'on conteste. à ce stade, en l'absence d'éléments vigoureusement cette estimation mais nous prenons acte de, de, de ce qu'elle l'emporte sur le sol budgétaire de l'État, telles qu'à ce moment, le gouvernement en fait l'estimation, Monsieur le Ministre, dans l'attente de la réunion de la commission mixte paritaire, nous proposons donc de supprimer ce dispositif qui a été voté en première délibération mais nous souhaitons nous précisons que nous souhaitons pouvoir trouver dans la la navette, un cadre pour permettent d'avoir un chiffrage qui puissent être partagées et je dirais accepter ce qui facilitera, convenons-en, mais j'en ai déjà beaucoup parlé tout à l'heure, nos travaux pour la suite. Merci, monsieur le Ministre. Oui c'est un avis favorable sur cet amendement, qui revient donc sur le sous-amendement que j'évoquais tout à l'heure, qui avait été adoptée sur le mécanisme de contribution sur la ronde infra-marginal, je le dis, c'était il y a le crois je crois cinq ou six jours que ce vote la nuit, de le le les services de Bercy ont le temps d'analyser cet amendement et de le chiffrer et quand on dit qu'il est chiffré à 6 milliards d'euros, c'est qu'il est vraiment chiffré à 6 milliards d'euros puisqu'ils relevaient les seuils à partir desquels on taxe les profits de 60 % donc avis favorable pour revenir là-dessus, mais encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, dans quelles conditions, ça c'était fait et donc je suis pas là en train de, de critiquer quoi que ce soit ou d'accabler quoique ce soit, je précise simplement, madame la présidente, qu'à l'issue de ce vote, il faudra une nouvelle suspension de séance pour qu'on puisse vous produire le nouvel article d'équilibre et le nouvel article liminaire, qui fait suite au vote de ces trois amendements, puisqu'avec le vote de ces trois amendements, il y a 8 milliards d'euros de recettes en plus pour l'État : 1 virgule 3 milliards d'euros de recettes en moins et donc au total 6 7 milliards d'euros de recettes supplémentaires, il faut qu'on les intègre pour refaire un article d'équilibre et un nouvel article liminaire, donc on demandera une courte suspension de séance mais service avait déjà commencé à travailler en parallèle évidemment sur la nouvelle mouture. Monsieur Beuchere pour explications de vote. minime, même président de pardon, mes chers collègues, monsieur le ministre, je me rappelle très bien de cet amendement de cette série tout amendement dans la nuit de samedi à dimanche, mais je me souviens aussi que vous aviez dit que vous même vous n'étiez pas très sûrs de la l'article de toute façon on été rédigé, votre amendement donc ici on est en train, enfin je veux dire on fait un amendement peut-être à à moins 6 milliards mais on comme on sait pas la taille de l'amendement et le le texte définitif que vous aurez, vous voyez bien qu'on est à 6 milliards sur quelque chose de très émouvant et donc tout cela convenant ensemble ça sera votre mouture définitive sans doute dans un 49 3 façon qui vaudra mais vous voyez bien que ce que nous avons fait par ces amendements. Y compris ceux qui n'ont pas été accepté. C'est de vous alerter sur le risque potentiel et on voit tout de suite comment un amendement pourtant bien travaillé, qui dira le contraire, surtout vu l'auteur. Que on va vite dans des excès dans un sens ou dans un autre et ce sera très sensible, très sensible pour l'ensemble de nos entreprises, donc il faudra bien travailler ensemble, voilà ce que je voulais vous dire donc évidemment je voterai. Comme tout le monde pour éviter réparer mais la sensibilité, elle sera chez vous dorénavant. Madame Lavarde, explications de vote. Oui merci madame la présidente, alors bien évidemment, j'ai aucune difficulté à ce qu'on remette au vote ce sous-amendement, par contre j'ai Monsieur le Ministre, une question à vous poser, comme l'a dit tout à l'heure monsieur de La Haye, il y a un effet de vases communicants entre les charges de service public de l'électricité et le rendement de la contribution sur la rente infra- marginal dont aujourd'hui si vous chiffrez cet amendement à 6 milliards qui concerné un tout petit nombre, enfin un sous-ensemble des entreprises taxées que vous le chiffrez à A6, permettez-moi de m'interroger sur le montant de 11 milliards que vous nous avez présenté samedi comme rendement de la contribution vendredi prochain dans cet hémicycle, nous allons débattre du programme 345 qui incluent les charges de service public de l'électricité, il me semble que nous devrions avoir connaissance de l'ensemble des coûts du chiffrage de manière à pouvoir si besoin recalibrer ce qui est fait sur le 345. Merci, cher collègue, le président Karoutchi pour explication de vote. je trouve que c'est quand même bon enfin on va le faire, on va suivre le rapporteur général, mais sincèrement, bon allez sur ce par exemple sur l'amendement succession on nous avait dit d'abord 3 milliards, puis 1 milliard 400 millions puis dans le document qu'on a eu, on a 2 milliards, bon, on voit bien que tout ça est approximatif que sur le sous-amendement de Christine Lavarde 6 milliards bon, vous auriez pu écrire 5, écrire 5, 7, donc on a un peu l'impression quand même que tout ça est et pas très très stricte, mais ma question n'est pas là, on va le voter, on va suivre le rapporteur général simplement Monsieur le Ministre, vous disposez du 49 3 on ne sait pas ce que vous allez faire, à l'Assemblée et on ne sait surtout pas ce que vous allez faire après l'assemblée est-ce que par exemple sur le bouclier énergétique des collectivités est-ce que sur un certain nombre de sujets qui concernent au 1er chef nos collectivités, vous pouvez au moins nous dire que ce qu'a fait le Sénat ne sera pas détricoter. Pour vous réponde, monsieur Karoutchi s'il y a bien un amendement pour lequel on a assez peu de doutes sur le chiffrage, c'est celui sur les droits de succession, c'est une mesure qui a été chiffré depuis longtemps parce qu'elle est dans le débat depuis longtemps, par ailleurs, nous nous sommes engagés à la mettre en oeuvre dans le courant du quinquennat donc je vous redis j'ai jamais parlé d'un virgule 4 milliards ces 2 milliards d'euros pour la partie état il y a 1 milliard pour la partie Sécu et c'est pour ça qu'on parle de 2 milliards d'euros avec le rapporteur général puisqu'on parle ici de la partie de la partie. Sur la 2ème question que vous posez, j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre le sens de la question puisque. Je peux non mais au moins sur une partie, ben non, mais parce qu'en fait, en fait, je vous semblez partir du principe qu'une fois que le budget aura été adopté à l'Assemblée nationale vous refuseriez qu'on l'examine à nouveau ici sur toutes les dimensions du texte je sais pas si vous avez déjà prévu de voter une question préalable pour le rejeter quand il reviendra, par définition, le le budget doit revenir ici ben donc quand vous me demandez : quand vous me demandez : que vont devenir les mesures qui ont été adoptés par le Sénat, on va revenir ici devant le Sénat, on aura l'occasion de revenir sur tous les articles

Je vais donc mettre aux voix cet amendement parce qu'il faut qu'on avance puisqu'après, nous avons l'émission, vous savez, chers collègues, et là nous sommes en train d'décaler gentiment vers le samedi donc je mets aux voix, c'est très important, je ne dis pas, mais je rappelle quand même, je rappelle quand même que je souhaite pouvoir mettre aux voix cet amendement avec de la commission avec un avis favorable du gouvernement qui vote pour. Qui vote contre. Qui s'abstient. Qui ne participent pas au vote, il est donc adopté. C'était une suppression d'alinéas je mets donc aux voix l'article IV du Ovi Siess ainsi modifié qui vote pour. Contre, abstention ne participe pas au vote. Il est adopté, nous en venons à l'article liminaire et à l'article d'équilibre, vous n'êtes pas donc en mesure de présenter dans l'instant, vous souhaitez une suspension de séance, vous savez à peu près le temps. Oui, alors l'article d'équilibre vient de vous être envoyé à l'instant, puisqu'on avait demandé, j'avais demandé qu'on le prépare en parallèle de nos débats en anticipant que les amendements seraient adoptés l'article liminaire est en cours de finalisation, on me dit que pour être séjour ou sur une quinzaine de minutes de suspension nous permettrait d'en d'en disposer dans les délais.

heures. Reprenons la séance chers collègues. Le tribunal. Nous passons donc à l'amendement du gouvernement sur l'article d'équilibre amendement numéro 5 Monsieur le Ministre, pour présentation. Merci madame la présidente, donc on tient compte du nouveau vote qui a eu lieu sur les 3 articles qui ont été supprimés, si je devais résumer les choses, je dirais que quand nous sommes arrivés dans cette assemblée, le projet de loi de finances prévoyait un déficit à 5 % conformément à la trajectoire que nous avons fixé 8 virgule 9 % en 2020, 6 5 en 2021 5 % cette année 5 % l'année prochaine et une trajectoire ensuite pour revenir sous les 3 % d'ici à 2027, au terme du première article d'équilibre et du de l'article liminaire que je vous ai présenté, on était passé suite au père. De de recettes qui avait été voté à 5 2 pour de déficit, vous avez adopté 3 amendements en seconde délibération de suppression d'articles pour revenir sur certaines pertes de recettes que je ne détaille pas, et nous sommes donc désormais avec un solde public à 4 9 % en très légère amélioration par rapport au à la copie que nous avions présenté à 5 % je précise que ce 0,1 point d'amélioration se fait exclusivement sur le dos, entre guillemets, des entreprises puisque il se fait grâce au fait qu'on ne supprime pas la CVAE si nous si vous aviez voté comme je l'aurais souhaité la suppression en deux fois de la CVAE le solde à l'issue de cet examen serait de 5 virgule 1 % donc en dégradation par rapport à la copie du gouvernement, je le redis, je regrette que. que je regrette que des centaines de milliers de PME de TI, notamment dans l'industrie au terme du vote qui a été effectué ici ne puissent pas bénéficier d'une baisse d'impôts de production l'an prochain, alors qu'on a un enjeu très fort de réindustrialisation, mais sur ce point, j'ai été assez clair sur le fait qu'on proposera évidemment en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, de rétablir la suppression de la CVAE en deux fois pourquoi est-ce que le fait d'avoir ses 4 milliards de recettes supplémentaires par rapport à la copie du gouvernement ne fais une amélioration que de 0,1 point parce qu'il reste un certain nombre d'amendements que vous avez adopté de pertes de recettes, il y a donc la nouvelle trajectoire sur la TGAP 133 millions d'euros, le relèvement du plafond de l'liesse PME pour le coup, là je le dis, qui bénéficie effectivement aux PME de 320 millions d'euros, l'amendement, garde d'enfants à 250 millions d'euros et 700 millions d'euros de baisses de TVA notamment sur la margarine sur les chevaux et sur les transports de voyageurs, donc je, je le dis, il y a, à l'issue de cette première partie. Un déficit à 4,9 j'ai noté dans la loi de programmation des finances publiques que vous aviez adopté que vous fixez un objectif de déficit pour 2023 à 4 6 ça veut dire qu'à l'issue de cette première partie, vous n'avez fait qu'un quart du chemin qu'il vous que vous devez faire pour arriver à un déficit de 4,6 ce qui veut dire que dans l'examen de la partie de de ce texte et les crédits budgétaires qui vont être examinées, il vous faudra trouver 10 milliards d'euros d'économies en net pour arriver, non, on vient de passer les recettes, donc là, on va passer dans les crédits, donc ça veut dire que vous allez devoir ponctionner, je parle à la majorité sénatoriale, évidemment, de 10 milliards d'euros les missions budgétaires que vous allez examiner dans les jours et les semaines à venir, je le dis vraiment sans aucune malice, j'ai hâte de voir parce que je suis très curieux, je suis très curieux, j'ai hâte de voir où est-ce que vous allez ponctionner 10 milliards d'euros est-ce que c'est sur la défense est-ce que c'est sur la sécurité est-ce que c'est sur l'environnement est-ce que c'est sur l'éducation nationale, il y a 10 milliards d'euros que vous allez devoir trouver dans la partie de pour être conforme aux objectifs que vous vous êtes vous-même. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Bon, d'abord, je, je veux dire que je prends acte des de la présentation qui a été faite par le ministre de l'article liminaire de l'article d'équilibre puisqu'ils résultent des votes auxquels nous avons procédé il y a quelques instants, il en tire les conséquences et donc dans la vérité des chiffres et du document présenté ce sera un avis favorable mais Monsieur le Ministre. Sans malice. Aucune. même pas cacher sans aucune perfidie non plus, vous évoquez l'objectif que nous avons que nous nous étions fixé de ramener déficit à 4 6 c'était en même temps, au même moment que vous aviez-vous comme inscrit dans le marbre comme objectif et 4 7 %. Donc pour le déficit 2023, je pense qu'à ce stade. Je ne suis pas sûr que les uns ou les autres, et vraiment de leçons de conduite et de respect des objectifs fixés à se donner, je m'en tiendrai là je crois que la situation, on l'a dit et difficile, mais vraiment je j'envoie un message je au nom de de de cette assemblée, c'est le la grande vigilance et le sérieux avec lequel nous allons continuer de travailler évidemment toute l'émission, mais vraiment sur les sujets d'énergie en se mettant à la fois à la place des consommateurs, où qu'il se trouve quelque que soit leur qualité, je leur ai dit qu'il soit particulier usagers soit des entreprises et associations et aussi et surtout vis-à-vis de nos acteurs économiques. Voilà que le message soit bien entendu et nous sommes disponibles pour être aux côtés de celles et ceux qui veulent travailler parce que, il va falloir plutôt se retrouvent, c'est les manches que de vouloir éventuellement sur ces sujets, profiter de difficultés des uns ou des autres. Merci monsieur Bocquet pour explication de vote. Oui, un petit commentaire avant de procéder au vote alors tout à l'heure, nous avons eu un petit mouvement d'humeur en ne participant pas délibérément au vote. Voilà, ça a été pris en compte et j'ai expliqué un peu les choses, vous parlez d'équilibre Monsieur le Ministre, mais quels équilibres de quel équilibre parle-t-on. On vient de nous proposer 3 amendements successifs pour rééquilibrer selon vos termes les choses mais on est en commission des finances, on est sur une loi de finances, qui doit être précise, précise, rigoureuse et voilà le libellé des amendements, alors je n'incrimine pas du tout notre rapporteur général qui a fait ce qu'il a pu, dans les circonstances qui lui ont été imposées, pas même que pas plus que la commission, mais on nous dit sur l'amendement numéro un, son coût pour les finances publiques s'élève de fait au minimum à plusieurs centaines de millions d'euros, c'est trois ce cette celui de ces quatre, on ne sait pas 2ème amendement. Le coût de l'amendement en question pour les finances publiques s'élèverait à environ 2 milliards d'euros environ, et le troisième même tonneau un coût pour les finances publiques d'environ 6 milliards d'euros, d'après le gouvernement, j'ai vraiment du mal à comprendre comment on peut voter de tels amendements et les soumettre au débat, ça fait huit jours qu'on est en discussion, et d'ailleurs, Monsieur le Ministre, je salue votre courage et votre capacité à répondre à tout le monde dans les débats qui ont eu lieu depuis 8 jours, vous vous dites attachée au débat, mais à l'Assemblée nationale, on a eu le 49 3 et au Sénat le 49 3 ne s'applique pas, mais on a la seconde délibération et le problème est réglé, il se passe des choses dans la coulisse, on a vécu une réunion de commission absolument lunaire tout à l'heure des passages de certains collègues, des coups de fil des conciliabules, des petits apartés et tout ça pour arriver au résultat d'aujourd'hui, franchement, ça n'est pas acceptable cette façon de traiter le Parlement était l'accepte pas nous la condamnons. Oui, moi, Monsieur le Ministre, je je voudrais revenir un instant sur votre déclaration à l'instant de présentation en disant en gros, les choses se font sur la base de de 4 milliards d'euros sur le dos des entreprises, avez-vous dit, c'est une curieuse façon de présenter les choses, pour plusieurs raisons : la première c'est que jusqu'à nouvel ordre, il y a rien pour l'instant, pour les entreprises, c'est au vote final éventuellement qu'il peut y avoir quelque chose, donc aujourd'hui nos délibérations ne sont pas sur le dos des entreprises mais je vous propose une formulation plus heureuse, c'est de dire, au bénéfice des citoyens, vous voyez c'est c'est autre chose, c'est une autre façon de voir, parce que de toute façon, ceux-ci ces 4 milliards, ils seront payés sur la dette, c'est-à-dire sur. La population d'une part et directement sur à travers la TVA par les citoyens non je crois qu'il faut être positif, cette façon de voir les choses, enfin vous avez très franchement et nous le savions que vous souhaitiez remettre suppression de c'est eux, dans le cas du 49 3, nous le savions, je voudrais juste rappeler que la première fonction du Parlement, c'est de voter l'impôt, la première historique depuis comme Parlement existe dans ce pays, sa fonction première, c'est de voter l'impôt à l'Assemblée nationale, refus au Sénat refus attention à ce que vous faites avec le Parlement monsieur le ministre. très très rapidement, monsieur le Président rénale je ne conteste en aucun cas la légitimité du Parlement, a décidé de revenir sur une baisse d'impôts que nous avons proposé. En aucun cas j'ai le droit de la regretter. J'ai le droit effectivement de considérer et de préférer, j'aurais préféré, parce que vous dites, c'est au bénéfice de la dette des déficits, le déficit ne bouge quasiment pas par rapport à la copie que nous avons, nous avions proposé au départ, on est à 4 9 par rapport à 5 % et donc s'il ne bouge quasiment parce parce qu'il y a d'autres pertes de recettes et j'assume de dire j'assume, je sais qu'il y a des secteurs qui sont aussi attentifs aux amendements que vous avez adopté j'assume de dire que j'aurais préféré qu'on baisse les impôts de production de 4 milliards d'euros, plutôt que la TVA sur la margarine, la TVA sur les chevaux, même si je sais que c'est très attendu par le secteur, on le fera je pense dans les prochaines années, la TGAP et d'autres mesures de perte de recettes que vous avez adopté voilà, je rappelle que la suppression de la CVAE estimé par la direction générale du Trésor à 150000 créations d'emplois dans les 3 années qui viennent, c'est des estimations mais en tout cas, on a vu avec les baisses d'impôts de production précédente que ça avait un impact, je voulais simplement répondre à monsieur Bouquet j'ai repris l'amendement du gouvernement, il est très précis. On dit sur les droits de mutation, les recettes sont dégradés de 2 milliards d'euros, compte tenu de l'amendement, on dit sur les l'assurance-vie améliorent les recettes de 1 milliard 300 millions d'euros, donc ce à quoi vous faites référence, ce ne sont pas des amendements du gouvernement, c'est les amendements de la commission d'on ne pouvait pas dire que c'est un manque de respect du gouvernement au Parlement, c'est pas nous qui avons fait les amendements et je les remets absolument pas en question, tout ça se fait de manière très rapide, mais je tenais quand même à le dire, il y a pas de conditionnel sur dans l'amendement du gouvernement sur les recettes et les dépenses. Merci, Monsieur le Ministre, je mets donc aux voix cet amendement sur l'article d'équilibre. Avec un avis favorable de la commission. Qui vote pour.

parfait, il est donc adopté, nous passons, monsieur le ministre à l'amendement article sur l'article liminaire amendement numéro 6. Je l'ai défendu avec le précédent. Avis de la commission favorable. Pas d'explication de vote je mets donc aux voix cette madame Lavarde. me laisse un peu dubitative à l'inverse, les recettes issues de l'extension de la contribution sur la rente marginal des producteurs au 2ème trimestre viendrait et de réduire le déficit public d'un peu plus d'un milliard donc un milliard pour 6 mois. Comment on trouve le des montants aussi élevé sur 2023 c'est, enfin c'est juste pour comprendre en fait. Monsieur le Ministre. il y avait notamment le fait que la taxe sur les superprofits que nous avons porté qui est issu du mécanisme européen devait démarrer au 1er décembre de cette année, j'ai proposé dans l'amendement que la taxe sur les superprofits des énergéticiens démarre non plus au 1er décembre mais au 1er juillet les Allemands la font démarrer au 1er septembre les pays choisis des dates différentes, c'est notamment pour nous, ce qui permet de rattraper les énergéticiens qui sont sortis du de la CSPE et donc ça ramènera ça rapportera un milliard d'euros effectivement sur 2022 de la faire démarrer au 1er juillet. Alors je je je rebondis, pardon, parce que, et pour le compte rendu ou ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas entendu la question de Christine Lavarde qui était pas au micro, elle dit un milliard sur 5 mois en 2022 comment est-ce que la taxe rapporte autant sur 23 parce qu'on est pas sur les mêmes prix sur les mêmes hypothèses de prix et donc forcément en 2023, on sait que les les les prix sur le marché de l'électricité seront plus élevés que ceux qui n'étaient a sur la période dont on parle en 2022, et donc que la taxe aura un rendement plus important. Alors j'ai mis aux voix, cet amendement avec un avis favorable de la commission qui vote pour.

Même vote, il est donc adopté avant de passer au vote sur l'ensemble de la première partie, je vais donner la parole à ceux de nos collègues qui ont été inscrits par les groupes politiques pour expliquer leur vote je rappelle au Sénat que conformément à l'article 42 de la loi organique relative au jour là de finances du premier août 2001 et à l'article 47 bis alinéa 2 de notre règlement lorsque le Sénat n'adopte pas la première partie du projet de loi de finances, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté, nous avons une estimation de 43 minutes de d'explication de vote, nous commençons par monsieur Rémi Féraud, du groupe socialiste, pour cinq minutes chers collègues.

Merci madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, chers collègues, c'est à nouveau dans un contexte exceptionnel que nous étudions cette année le budget de l'État, sorti de la crise sanitaire, prolongé par une autre crise inflationniste due à la guerre aux portes de l'Europe, remontée des taux d'intérêt menace de récession et inquiétude sur l'avenir, mais nous l'étudions aussi dans un contexte qui voit de grandes tendances contradictoires marqué profondément l'évolution de notre société, d'un côté des profits toujours plus important des grandes entreprises avec des dividendes versés, qui ont un niveau atteint un niveau record, pas besoin de citer à nouveau les chiffres et de l'autre côté, une explosion de la pauvreté qui devraient nous mobiliser bien davantage le Secours catholique, comme les Restos du Coeur dresse d'ailleurs un constat sans appel, le nombre de leurs bénéficiaires augmente et leurs difficultés également, bref, les riches n'ont jamais été aussi riches et les pauvres aussi pauvres or que propose le budget de ce gouvernement pour enrayer cette dynamique qui voit les inégalités s'aggraver toujours davantage. Rien sur la taxation des superdividendes et si peu sur la taxation des superprofits dont nous avons pourtant longuement débattu ici d'autres pays européens ont mis en place une contribution exceptionnelle, sans atteindre sans attendre celle voulue par l'Union européenne pour les seuls énergéticien la France non, et le Sénat n'a malheureusement pas changer cela, rien sur le rééquilibrage de la fiscalité, le gouvernement continue de baisser les impôts de production de ménager les plus fortunés de refuser la création d'un ISF climatique alors que l'échec de la politique du ruissellement n'est plus un secret pour personne, dans son rapport, le FMI lui-même, remet en cause la pertinence de cette politique en ce qu'elle participe activement du maintien d'un déficit public trop élevé dans ce budget, rien non plus de durable pour le pouvoir d'achat des plus modestes, rien à la hauteur de cette inflation qui les appauvrit en 1er lieu ristourne temporaire aide ponctuelle, le gouvernement s'en-tête à refuser toute mesure structurelle qui aiderait réellement nos concitoyens les plus en difficulté, à commencer par une grande conférence sur les salaires par la politique fiscale qui est menée et qui protège les plus aisés et les grandes entreprises, vous ne vous donner de toute façon pas monsieur le ministre, a les moyens d'une meilleure redistribution et les réformes que vous engagez vont même aggravé la situation réforme des retraites, bien sûr, mais dès à présent, réforme de l'assurance chômage pour trouver de l'argent, vous préférez taxer les chômeurs que les super profits et le déséquilibre qui caractérisait votre politique lors du premier quinquennat se poursuit avec l'approbation de la majorité sénatoriale dont on a bien senti tout au long des débats que le budget présenté lui convient en réalité sur les points essentiels ensemble vous persistez dans cette politique économique et fiscale en faveur du capital alors qu'elle devrait avoir de priorité le travail et le climat, enfin je veux avant de conclure : revenir sur l'enjeu essentiel des collectivités territoriales après la taxe d'habitation, le gouvernement s'attaque cette année à une autre ressource la CVAE, la méthode est la conséquence restent les mêmes : dès que vous acter une baisse d'impôts, l'État s'appauvrit en perdant des recettes de TVA et les collectivités territoriales aussi car elles sont la variable d'ajustement, cependant, et contre l'avis du gouvernement, nous avons fait des progrès notables dans la discussion au Sénat et disons-le aussi clairement des progrès souvent arrachés à la majorité sénatoriale, c'est un autre initiative notamment que nous avons eu la sagesse de d'annuler la suppression de la CVAE, je m'en réjouis, nous avons aussi voté l'indexation de la DGF sur l'inflation, comme nous le proposions et améliorer le filet de sécurité pour les collectivités, grâce à ses votes le Sénat montre qu'il est et qu'il reste la chambre qui défend les territoires qu'en restera-t-il 49 3 ou pas au gouvernement maintenant de prendre ses responsabilités et de les assumer devant les devant les élus locaux et nos concitoyens. Mes chers collègues, nos votes favorables aux collectivités ne bouleverse cependant pas le déséquilibre profond d'un budget que nous considérons comme injuste et imprévoyant, les chiffres de l'Insee ont montré cette semaine que les 2 dernières années ont été favorables aux plus riches de nos concitoyens, je vous l'annonce, avec ce budget l'année prochaine le sera également, alors le groupe socialiste, écologiste et républicain votera évidemment contre cette première partie du projet de loi de finances, je vous remercie.

Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues. Qu'est-ce que provoquer. C'est à avoir le courage d'affronter des idées reçues et de s'opposer à la pensée majoritaire, c'est pas de moi, c'est Élisabeth Badinter. Par le dépôt d'une question préalable, nous étions opposés par la voix de notre présidente. Le groupe CRCE exprimé les craintes sur les conditions politiques du gouvernement, rendant le débat et ça s'est vérifié menacée. Le débat a été faussé mais aussi sous l'arbitrage des droites du Sénat, on vient de le voir il y a encore quelques minutes avec 3 amendements ou le Sénat s'excuse, baisse la tête en disant : je me suis trompé dont tac le gouvernement, il faut faire attention et puis après on est la suite, on a eu la la on a eu un petit moment de navette, je vous ai dit d'arrêter avec la navette, le ministre de la vérité avec la navette dont acte, mais là tout à l'heure qu'est-ce que vous nous dites-vous nous menacer. Attendez, ce que vous avez décidé et voté, faites gaffe, hein, il va falloir trouver 10 milliards de dépenses publiques en moins, donc c'est un 49 3 ça, enfin, ça s'appelle pas comme ça, constitutionnellement, mais c'en est un, politiquement, hé bien nos comportements, moi je vous le dis nos amendements ont été ceux d'une opposition politique de gauche au choix budgétaires du gouvernement et sur l'invocation de 4 49 3 sur les lois de finances de l'État, des collectivités et de la sécurité sociale depuis il y a eu un 5ème passage en force qui a eu lieu la démocratie parlementaire est encore une fois malmené, d'autres démocraties qui, pourtant, pourtant, devrait révéler toute sa promesse en cas d'absence de majorité. S'apparente à une succession de coups de butoir un coup sur le pop un coup sur ses aspirations et puis en même temps dans la foulée, ce ça représentant, il suffisait d'entendre le mot répété d'innombrables fois, tantôt laconiquement par vous. Tantôt après des tirades libéral, des fois, vous le savez, moralisatrice. Mais toujours conclu par défavorable. Les débats qui sont tenus sous le joug du 49 3 dans la ligne de mire d'un gouvernement défavorable par principe oppositions aux propositions, responsable des oppositions. Seul Ministre, mes chers collègues. C'est certes les les erreurs font partie de la vie, mais c'est la réponse qu'on leur oppose qui est importante : le Sénat vote et nous en fit, citons le maintien de la cotisation sur la valeur des entreprises plutôt que d'acter que la seule assemblée ayant pu débattent rejette la disparition de cet impôt, en se gardant bien de rappeler que les élus locaux étaient farouchement attachés à la territorialisation de la valeur ajoutée à ce lien économique entre la commune et le lieu de production, la CVAE n'est pas tant décrié par les entreprises elles-mêmes. Qui, n'en déplaise à je sais pas qui, ici, les entreprises, des chefs d'entreprise focalise sur quoi les infrastructures, la qualité du bassin d'emploi et du réseau de service, enfin, une aberration pour une France considérée par votre collègue, le ministre Lemaire, je le cite, à l'euro près. Il est à l'euro près tellement à l'Euro près que quand il faut passer outre le débat parlementaire, mais qu'il entend faire voter 9 milliards d'euros de baisses de CVAE pérenne, bonjour l'euro près et tout, et touche le concédait ce n'était ni possible, la Cour des comptes, le rappelait, ni le moment ni souhaitable, il arrive que nous votions la même chose ici, il est plus rare que ça soit pour les mêmes raisons, mes chers collègues, la clarté, la responsabilité m'invite à vous le dire, nous sommes pour la préservation et le renfort de la fiscalité économique territoriale pour une refonte du solde au plafond de la fiscalité des entreprises, monsieur le ministre, il nous faudra respecter ce vote, nous vous le demandons avec solennité respecter ce vote cette décision souveraine engage notre pays et elle vous engage. J'aimerais dire un mot sur un amendement adopté et cusez moi le le mot et respectueux mais ce je pense à un amendement scélérat. Le même amendement que celui adopté ici a été retiré par le gouvernement, juste avant la séance, il fallait protéger le ministre, l'Élysée avait décidé. Alors on utilise et sénateurs de la majorité en en marche renaissance enfin gouvernementale allez c'est plus, je veux pas vous ne veut pas, je sais pas comment, vous, des fois vous identifier, c'est plus discret, c'est moins engageant et c'est peu dire ça aidera les grandes entreprises, elles sont les seules à s'assurer elles-mêmes, via une filiale, ce qui constitue un outil d'optimisation des plus agressifs, les captives de réassurances sont pour la plupart hébergés au Luxembourg, en raison d'une fiscalité attractive version euphémisé de paradis fiscal au coeur de l'Europe, il est donc rendu non imposables provision auprès d'une filiale en prévision de tous les dommages de biens professionnels agricoles Caracas catastrophe naturelle, responsabilité civile et j'en passe, en gros ce qui vient de se faire, c'est on passe par-dessous pour faire un cadeau pour les plus grandes entreprises, c'est un non-sens économique, c'est la preuve d'un capitalisme qui aujourd'hui considèrent que toutes les marchandises et y compris Monsieur le Ministre, même le travail devient une marchandise, il a été force d'idée comme d'autres de persuasion en faveur des avancées majeures pour les collectivités territoriales, l'indexation de la DGF sur l'inflation, même si vous nous aurions préfère une indexation pérenne la compensation, département de la revalorisation du RSA sur l'inflation, l'engagement de la réforme de révision des valeurs locatives des locaux d'habitation ou encore l'intégration de la compensation de TVA, mais pour toutes les raisons que j'ai expliqué au tout début et le fait que, malheureusement, s'il y a bien des gens rassuré, c'est ceux qui font des superprofits et des profits, nous voterons contre cette loi, merci de votre attention. Merci, je passe la parole à présent Madame Sylvie Vermeillet, du groupe Union centriste pour cinq minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, avant de voter solennellement sur la partie recettes de ce 1er budget de la législature, je voudrais revenir un instant sur les grandes orientations qui le fixe et sur les points de vigilance du groupe Union centriste nous avons consacré les précédente loi de finances initiale et loi de finances rectificative au sauvetage de notre économie face à la crise sanitaire et l'examen de ce projet de budget pour 2023 a débuté au lendemain de l'adoption par notre haute assemblée d'un second collectif budgétaire 2022 lui-même destiné à protéger les Français face au danger qui que font peser l'ensemble de l'inflation élevée et la guerre en Ukraine et les aléas climatiques dépenses dépassant de beaucoup la conjoncture immédiate, la succession de ces crises mais lourdement à contribution nos finances publiques. Or le resserrement de la politique monétaire amorcé par la Banque centrale européenne pour juguler l'inflation change inéluctablement la donne budgétaire dans ces conditions, certes nouvelle mais néanmoins attendu les membres du groupe Union centriste, aborder ce projet de budget 2023 dans un esprit de responsabilité fidèles à notre ligne constructive nous avons été, force de proposition, oui nous devons collectivement concourir au redressement des comptes publics afin de conserver la maîtrise de notre destin, notre groupe juge néanmoins impératif d'associer à la maîtrise des dépenses publiques, l'optimisation des rentrées fiscales dans les caisses de l'État. En votant la suppression de l'article 5 nous avons voté le maintien, pour l'année 2023 de 4 milliards d'euros de CVAE aujourd'hui perçue par le bloc communal et les départements, l'objectif affiché n'est pas seulement de préserver l'autonomie financière des collectivités locales, il est aussi de sauvegarder les substantielles ressources publiques dont on ne peut se priver pour financer les soutiens exceptionnel aux entreprises, nous avons également concrétisées dans ce projet de budget plusieurs propositions volontaristes visant à rationaliser notre système fiscal dans un double souci d'efficacité économique et d'équité sociale, le remplacement de l'impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive je songe aussi à la suppression d'une niche fiscale implicite sur la transmission du Patrimoine des plus fortunés qui contournent l'impôt sur le revenu en exploitant une faille du nouveau plan d'épargne retraite, issu de la loi pacte en faisant adopter notre amendement nous avons corrigé une anomalie qui se chiffreraient d'après certaines à plusieurs plusieurs milliards, mais qui n'est pas évalué dans l'article d'équilibre qui nous a été présenté. Nous nous réjouissons par ailleurs des parvenu avec le concours et l'aval du rapporteur général de la commission des finances, à améliorer et renforcer le dispositif de filet de sécurité en faveur des collectivités territoriales, monsieur le Ministre, les élus du bloc communal confrontée à l'explosion de leurs dépenses d'approvisionnement en énergie ont besoin d'une réponse claire lisible et rapide, nous espérons vivement que le dispositif adopté par le Sénat survivra au 49 3. Voilà un bal à un balayage nécessaire rapide et non exhaustif des apports du Sénat et de notre groupe que nous voulions mettre en valeur avant le vote solennel qui aura lieu dans quelques minutes monsieur le Ministre, je vous ai entendu il y a quelques instants, nous a signé une trajectoire d'économie pour la seconde partie du budget, je vais tout de même vous rappeler que nous venons depuis 8 jours ne vous proposer des milliards de recettes supplémentaires et des milliards de suppression de dépenses fiscales parce qu'elles ne vous conviennent pas, vous les ignorez le groupe Union centriste est allée bien au-delà du redressement attendu et je vous prierai de l'entendre, bien évidemment, nous regrettons de ne pas avoir pu élargir la contribution exceptionnelle de solidarité à l'ensemble des secteurs d'activité économique, au-delà du seul secteur de l'énergie, il demeure inacceptable de taxer certains sans limite, particulièrement ceux qui ont besoin de ressources pour réussir leur transition écologique, quand d'autres, non concernés continue d'accumuler des profits records cette obstination à instaurer des privilèges dans un contexte de déficit public bien trop excessif. Engage la responsabilité du gouvernement mais 2023 ne nous a encore pas tout dit, et peut-être que nous n'auront plus le choix, dans quelques mois, quoi qu'il en soit, mes chers collègues, le groupe Union centriste salue la qualité des échanges que nous avons eu dans cet hémicycle et continuera à être force de propositions pour la suite de l'examen du PLF nous voterons en faveur de la première partie du projet de loi de finances pour 2023 je vous remercie. Merci, cher collègue chapelle là présent Monsieur Christian Billac. Pour le groupe RDSE, vous avez 5 minutes chers collègues. Madame la présidente, monsieur le Ministre ça, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. à l'issue de la première partie du projet de loi de finances pour 2023, l'heure est à la fois la prospective au bilan après un budget de Milové NT1 sous le signe du Covid budget 2022 sous le signe de allais action : le budget 2023 s'inscrit sous le film et le bouclier énergétique et d'une inflation qui s'installe, je me permettrez d'abord de rappeler que l'année dernière, notre débat budgétaire avait été tronquée par le rejet de la première partie, par une majorité sénatoriale. jours confidence : nous avons été privés, ainsi de la 2ème partie de la discussion budgétaire, le groupe RDSE avait voté en faveur de la première partie, non pas pour approuver ce document mais pour permettre la poursuite de la discussion et conforter le rôle du Sénat et le BK auquel notre groupe est très attaché, c'est pourquoi je me réjouis que cette année, la discussion budgétaire aille à son terme, elle est marquée par un fil directeur : la prise en compte du contexte énergétique inflationniste pour les particuliers pour les entreprises et pour les acquéreurs, l'activité locale si je regrette la réduction de notre dette toujours abyssal et qui est reportée à des temps meilleurs, je comprends aussi la volonté du gouvernement de répondre aux demandes et aux inquiétudes. Les questions portant sur la taxation des profits, l'impôt sur le revenu et la redistribution ont occupé les débats du Sénat, tout comme celle sur la fiscalité, un autre maire autour de la mode de mal entre collègues, Stéphane Artano dirais pour ma part déposé 2 amendements qui n'ont pas été adopté, je le regrette, si je me félicite que le Sénat est rendue facultative le partage de la taxe d'aménagement entre les communes, les intercommunalités, je regrette que bon d'devant un restaurant le paiement de cette taxe à l'ouverture du chantier plutôt qu'à la déclaration d'achat aux mains des travaux n'ait pas été retenue, cela va plonger dans beaucoup de collectivités et de particuliers dans des difficultés financières, dont nous reparlerons autre regret mon amende globale sur le report de la révision de voir locatives pour les locaux d'habitation n'a pas été retenu, je continue de penser que, face aux difficultés et aux incohérences constatées dans la révision de locaux professionnels, c'est une erreur de continuer avec le même canevas, il aurait fallu en tirer les conclusions et c'est beaucoup plus de liberté de manoeuvre aux commission communale des impôts Directs, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on risque d'arriver rapidement à un constat d'échec, je regrette aussi. Le rejet de nombreux amendements déposés par mon groupe RDSE mais ces remarques étant faites, je me réjouis que de nombreux amendements favorables aux collectivités territoriales trouver avait été adoptée, et je tiens à évoquer tout particulièrement mal d'alignement de la Duchère sur l'inflation, ainsi que les mesures relatives à la TSR est favorable donc à la ruralité, à l'occasion des précédentes discussions budgétaires j'avais déposé des amendes de vidant des amendements visant à rééquilibrer modestement en faveur des territoires ruraux, la péréquation mises en oeuvre au moyen de l'ADSL, le texte de gouvernement va dans ce sens et au-delà de mes demandes en accordant 200 millions d'euros supplémentaires à la DSR, contre 90 pour la dotation urbaine et 30 millions pour la dotation d'intercommunalité, le critère de répartition d'EADS et as le Maroc était redéfini avec la mise en place d'une une dictateur prenant en compte la superficie la densité et la population, pour ma part je crois tu ne veux penser que le critère voirie était le meilleur mais je retiendrai l'effort fait pour la pluralité qui tend à réduire l'écart entre la DSR et la DSU, on commence à comprendre comme des champs doit autant être comme pauvres des villes, mais il reste encore du chemin à parcourir, je me félicite également que le portail dans les étaient supprimés pour l'attribution de la dotation élu local. Concernant le FCTVA je retiendrai l'amendement qui permet aux collectivités doivent bénéficier à nouveau pour les acquisitions et aménagement de terrains mais aussi pour les travaux, un régime après ce rapide panorama dans le temps, qui même parti je voterai donc favorablement pour ma part, en espérant que les travaux du Sénat soit pris en compte dans la version définitive et que la CMP sur le projet de loi de finances pour 2 matches de vingt-trois se tient dans le même esprit que celle du 2ème, projet de loi de finances dresse explicative pour 2022, que nous examinerons demain les membres du groupe RDSE se prononceront majoritairement en faveur de ce projet de loi en attendant la fin de la discussion budgétaire le remercie. Vous avez 5 minutes chers collègues. Merci madame la présidente, alors mes chers collègues, avant de commencer, moi je voudrais adresser des félicitations au rapporteur général et au Ministre qui viennent. Quand même de réussir une épreuve physique importante, qu'on n'avait jamais connu jusque-là. J'ai compté, nous avons siégé cinquante-sept heures sur cette première partie, alors Monsieur le Ministre, je vous invite à venir courir un semi-marathon dimanche en limite de votre circonscription, je ne sais pas si la performance sera au rendez-vous mais en tout cas, on aura l'endurance alors une fois ses bons mots passer et comme j'ai quelques doutes sur les conclusions de la CMP et comme Noël n'est pas si loin, j'ai envie de vous faire une sorte de petite liste sur les sujets qu'on apportés et qui nous semble vraiment important de conserver dans l'intérêt national, national, alors déjà, nous avons porté un certain nombre de mesures qui ont été adoptés, de soutien aux entreprises et notamment aux plus petites d'entre elles, les PME et je pense notamment ici, à la revalorisation du plafond du plafond IS pour les PME, nous avons aussi demandé que le bouclier que le filet de sécurité soit potentiellement accessible à toutes les communes, et nous le redisons ici introduire des critères, que ce soit la richesse l'épargne sont des critères qui n'ont pas de sens quand on vit un choc, un choc inflationniste d'une telle ampleur, je pense qu'on vous a proposé un dispositif juste en ce sens qu'il vient, permettre de laisser une un pourcentage de recettes pour financer le les autres choc inflationniste, le point d'indice, l'alimentation ou autre et venir apporter un soutien de l'État à toutes ces communes. Il nous semble aussi que pour pouvoir relancer l'investissement local, ce qui est particulièrement important, cette période et je rappelle ici que le 1er film, investisseurs, ce n'est pas l'État, mais ce sont les collectivités locales, il faut réintégrer dans l'enveloppe du FCTVA les dépenses d'aménagement de terrain, sans cela, ce sont un très grand un très grand nombre de communes, et notamment les plus petites, qui ne pourront plus faire vivre les les entreprises locales pour venir financer un aménagement de sites hier un terrain de foot, enfin, nous en avons largement débattu sur ces bancs, enfin et avant d'attaquer la seconde partie, je voudrais revenir sur mes propos de tout à l'heure, il y a tout un tas de sujets et notamment le sujet de l'énergie, nous savions que vous saviez que ce sujet serait au coeur du PLF, on a besoin d'avoir le même niveau d'information, sinon à travers la représentation, c'est aussi les Français qui sont un peu floués, où on leur cache des choses et j'avoue que, plus je vous entends plus une nouvelle question à vous poser, alors tout à l'heure, vous nous avez attaqué sur notre crédibilité au regard de la LPFP enfin, nous, on n'a pas la possibilité de sortir des nouveaux milliards des recettes imprévues imprévues ou autre, enfin voilà, aujourd'hui vous nous annoncez un montant de de de contributions sur la rente infra-marginal au regard de ça, moi je le mets sur les montants qui sont annoncées pour les amortisseurs si on attend sur la contribution, ça veut dire qu'il va falloir mettre plus sur les amortisseurs, sinon le dispositif ne marche pas, ou ça veut dire qu'on va avoir un certain nombre d'acteurs économiques qui vont se trouver en très grande difficulté l'année prochaine, alors je sais vous auriez envie de m'inviter un groupe de travail, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps d'ici vendredi prochain, mais j'ai noté en tout cas que ici, nous allons avoir un certain nombre de sujets à continuer à travailler ensemble, mais je me demande d'ailleurs s'il faut pas qu'on commence dès le 1er janvier parce que bien évidemment il va falloir faire un groupe de travail pour parler de la réforme des valeurs locatives et s'engager des à présent dans celle des, des, des valeurs locatives d'habitation et ne pas reporter ce sujet sans cesse, et surtout pas à 2025 très mauvaise année pour engager une telle réforme, nous allons aussi travailler sur le financement des transports alors en Île-de-France, ça sera de nouveau l'objet de débats dans la seconde partie, mais hier les amendements qui ont été déposées, montres que ce problème va bien au-delà du sel, le périmètre de la région Île-de-France et que cette question doit être posée et cette question, elle part, elle à la décarbonation de notre économie et à la transition écologique à laquelle vous aspirez à laquelle nous aspirons, il va peut-être falloir aussi faire un débat sur le fond Vert parce que on ne connaissait pas grand chose, mais la pluie, on en entend parler, plus on a l'impression que c'est le ramassis de tout ce qu'on n'arrive plus à financer ailleurs, donc nous aurons de nouveau ce débat, vendredi prochain, dans cet hémicycle et surtout et avant tout, mais il va falloir se mettre tout de suite sur la table pour travailler sur les modalités de compensation de la suppression de la CVAE pour les collectivités, parce que je le redis ici, notre groupe est très attaché à la baisse des impôts, de production, la seule chose qui nous a heurtés et pourquoi nous ne pouvions pas adopté l'article telle qu'il était proposé par le gouvernement, c'est que nous n'avions absolument aucune information, aucune garantie sur le fait que les modalités de compensation pour les collectivités, permettrait d'assurer un dynamisme et là vous voyez, Monsieur le Ministre, si nous avions eu ces groupes de travail avant de commencer à discuter, nous aurions peut-être pu trouver un accord à avoir un texte qui aurait pu permettre de concilier à la fois la baisse des impôts de production pour les collectivités, et en même temps d'assurer aux collectivités dans la durée, un maintien de leur dynamisme de recettes économiques, on a envie, à l'issue de cette première partie de vous inviter à continuer à travailler avec nous et surtout à nous donner plus d'informations pour qu'il ait le même niveau d'information, le même niveau de connaissances au moment où nous légiférons. Merci, cher collègue, la parole est à présent à notre collègue. Sénateur Emmanuel qui appuie pour le groupe des indépendants, vous avez 5 minutes, chers collègues, Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, l'objectif de ce budget, particulièrement cette année, c'est de rassurer les Français, rassurer les Français sur notre solidarité face à l'inflation, rassurer les Français sur notre volonté de tenir le cap, malgré les incertitudes liées à la crise en Ukraine et rassurer les Français sur notre sérieux budgétaire, il faut faire tout cela à la fois, mais l'urgence, cette année, c'est d'abord de maîtriser les coûts de l'énergie. Leur hausse menace la stabilité de notre économie. Nous avons à cette fin, voter des mécanismes de soutien face à l'inflation, le Sénat, les a drastiquement renforcée pour les collectivités en supprimant même tous critères d'éligibilité au filet de sécurité, en l'espèce l'amendement du rapporteur général sur l'article 14 nécessairement coûteux, même si j'ai remarqué que et j'ai bien compris que son impact n'étaient pas chiffrée dans l'article liminaire. Parce qu'il transfère aux collectivités et que du coup ça déséquilibre pas le le le le le l'ensemble, ce qui me paraît être quand même problématique sur le coût global. Elle est la bienvenue, cette évidemment, cet investissement est le bienvenu pour nos collectivités qui feront encore face à des hausses spectaculaires en 2023 je crois cependant, comme je l'ai dit, au cours de nos débats qu'il conviendra de mieux cibler ce dispositif et ce d'autant plus que le Sénat a déjà choisi d'indexer la DGF sur l'inflation, contre cette fois-ci l'avis de la Commission et du gouvernement. Pour préserver l'efficacité de nos dépenses, mes chers collègues, il conviendra nécessairement de retravailler ses critères d'éligibilité des critères d'éligibilité, simple et souple. Ces mesures de protection supplémentaires sont en partie financées par des recettes nouvelles obtenues notamment en taxant les super-profits liés à la hausse des coûts de l'énergie, ces recettes étaient pertinentes car elles sont bien calibrées, d'abord parce qu'elles sont européennes et non franco-française, ensuite parce qu'elle ne concerne que le secteur de l'énergie, précisément là où l'inflation prend racine. Je me réjouis que nous ayons résister à la tentation de taxer les super-dividendes culpabiliser les profits fustige réalisé en période de crise n'a jamais mené à la prospérité, mes chers collègues, Churchill considérait que le vrai vie ce sont les pertes non pas les profits je partage cet avis : il faut cesser d'inverser les valeurs. Rassurer les Français, c'est aussi leur montrer que nous gardons le cap malgré les turbulences, c'est notamment le cas pour la transition écologique cette priorité ne saurait être mise au second plan au motif que la crise frappe lourdement le Sénat a d'ailleurs renforcé l'ambition écologique de ce budget par des mesures concrètes et opérationnelles ne feront peut-être pas les gros titres, elle ne feront pas le besoin, en cela, elles sont très sénatorial mais elles font évoluer les choses dans le bon sens et c'est heureux, nous devons montrer aux Français que l'écologie, ce n'est pas jeté de la soupe sur des tableaux mais bien appliquer des solutions concrètes pour diminuer notre impact carbone. 2 amendements ont été ainsi adopté qui reprennent un texte porté par notre collègue Vanina Paoli-Gagin et le groupe des indépendants dans notre espace réservé, il vise à mobiliser davantage de fonds privés pour l'entretien de nos forêts, grâce au dispositif mécénat. Je m'en réjouis, en résumé, mes chers collègues, malgré des avancées positives, nous avons un regret qui brouille le message ce regret porte sur la CVAE, notre groupe a défendu une ligne claire supprimer cet impôt qui plombe nos entreprises et compenser les collectivités à l'Euro près de façon dynamique et territorialisées. Les élus locaux sont inquiets et nous devons le le leur assurer qu'il n'y perdront pas d'abord parce qu'en renforçant la compétitivité, on soutient les collectivités, ensuite parce que la TVA demeure la recette la plus sûre en temps de crise, surtout, même en temps de crise. Si les forces du centre et de la droite s'accordent et Christine Lavarde, la rappeler pour dire que la CEVA n'est pas un bon impôt, alors nous devons collectivement à avoir le courage de le supprimer. Définitivement. Mais proposer un report puis voté un dégrèvement et enfin ne pas voter l'article du tout, il me semble que ces mortiers de clarté vis-à-vis des élus locaux, de ce point de vue, je regrette monsieur le rapporteur général qu'il n'y a pas eu de seconde délibération sur la CVAE. C'est un regret. Il me semble qu'il y a une majorité qui partage mon avis et notre avis sur ce ce dispositif en tout état cause notre gros bout l'arrêt peut être compris et en tous les cas, si vous ne l'avez pas compris, je vous le précise s'abstiendra dans sa majorité sur cette première partie et pour quelques-uns la votera. Je vous remercie, la parole est à présent notre collègue Daniel Breuiller du groupe écologiste, vous avez 5 minutes chers collègues. Madame la présidente, monsieur le rapporteur général, monsieur le président de la Commission, monsieur le Ministre, d'abord, félicitations à à vous tous pour la tenue de ces débats et Monsieur le Ministre, pour votre implication, pas pour les avis que vous avez rendu mais en tous les cas pour vos réponses à nos interrogations au début de nos débats j'avais interrogé la sincérité du gouvernement et l'utilité de notre travail, sous la menace du 49 3, je dois dire qu'à l'issue, je doute toujours de la volonté du gouvernement de prendre en compte les débats et les décisions, les amendements votés au sein de notre assemblée, nous sommes entrés dans ce débat avec un cadre posé par le gouvernement, qui mettait les collectivités sous tutelle et refusait de demander toute contribution supplémentaire à ceux qui accumulent richesse et profits refus validé et même renforcé par notre rapporteur général et le groupe majoritaire du Sénat et puis le Sénat a débattu de façon authentique, parfois, la vie est même entré avec force, celle des territoires bien sûr et celle des habitants de notre pays, pour répondre à la volonté de diminuer le déficit et de renforcer les moyens de l'État, vous aviez une solution taxer ceux qui profitent de la crise qui vivent non de leur esprit entreprenarial, mais d'une rente générée par cette crise ou taxer les énergéticiens mais pas les super profits de l'énergie carbonée de la pharmacie du transport maritime ou de la banque et bien sûr pas non plus les dividendes, les centristes proposait de taxer les dividendes à la hauteur de la fiscalité du travail quand on prétend défendre la valeur travail, cela ne me semble pas scandaleux, ça n'était pas non plus avant le la nuit du 4 août je suis élu d'une commune populaire mes compatriotes qui vont aux distributions alimentaires ne comprennent pas que l'on ne taxe pas ces super profits alors que nous n'avons pas les moyens de nos politiques sociales, anticipant cette colère sourde comment les Françaises et les Français qui ne cesse de se débattre pour savoir comment se chauffer, se soigner, se déplacer et vivre bien peuvent-ils comprendre que la rémunération moyenne des patrons du CAC 40 représente cent neuf fois celle de leurs salariés, ce texte ressort sur plusieurs aspects plus dur socialement qu'ils ne l'étaient à l'origine, fruit là aussi de la majorité sénatoriale qui vous concurrence Monsieur le Ministre, dans le toujours plus libéral sur la CVAE, bonne nouvelle pour notre groupe, la suppression de la CVAE aurait été une erreur et même une faute que de priver l'État de 8 milliards d'euros de recettes, je m'étonne là encore que la majorité sénatoriale soutiennent la suppression d'un impôt qui lie les entreprises au territoire et qui finance les collectivités territoriales, la compensation par la TVA, taxe la plus socialement injuste va transférer un impôt des entreprises sur le dos des ménages respecte Trévoux, Monsieur le Ministre de la décision du Sénat. Pour la dotation globale de fonctionnement, une majorité très large s'est exprimé pour son indexation sur le taux d'inflation exigence aussi pour préserver les collectivités avec un filet de sécurité renforcée, mais là encore, notre vote sera-t-il respecté au vu de vos déclarations, vous semblez tenir pour acquis que non, vous pensez à voix haute, votre choix de 49 3 Izé nos votes et amendements, les débats que nous avons eu sur le logement, et plus particulièrement sur le logement social ont fait renaître une colère qui m'animait lorsque j'étais maire, l'objectif du gouvernement de construire 250000 logements est loin d'être atteint des dizaines de milliers de familles sont mal logées, la pénurie de logements n'a jamais été aussi importante, la fondation, la Fondation Abbé Pierre nous alertent le Secours populaire a vu le nombre de personnes a aider augmenté de 45 % notre débat et surtout ses conclusions n'ont pas été à la hauteur de ces enjeux ni des souffrances sociales générées par le mal logement, chacun a besoin de l'autre, avez-vous dit monsieur le ministre et conseiller municipal, c'est vrai, alors respecter les mesures votées dans cet hémicycle en faveur des collectivités, les prix augmentent l'inflation frappe d'abord les couches moyennes et les gens les plus modestes et les Français en difficulté se tournent vers leur mère qui doivent avoir les moyens d'agir pour les écologistes, mais surtout pour la transition écologique, le nombre d'amendements adoptés et plus que décevant, on a entendu fond Vert, fond Vert, fond vers 2 milliards recyclé puis qui devait tout résoudre, mais notre déception n'ni rien, l'incapacité à prendre la mesure de la crise climatique et tout, beaucoup de nos concitoyens de nos enfants, de nos petits-enfants ne croit plus en nous les politiques, pour ces raisons, pour notre incapacité à faire face à cette crise qui grandit et nous menace tous, beaucoup de nos propositions vous paraissent trop trop fort, trop rapide, trop mais si nous ne nous engageons pas rapidement dans cette trajectoire de transition, il sera vite trop tard, l'écologie n'est pas un dogme, c'est une nécessité, avec l'exigence de justice sociale, c'est même la trajectoire d'avenir de notre pays et de notre planète, c'est pourquoi nous ne voterons pas cette première partie de budget. Si cher collègue, enfin j'appelle. Pour explication de vote, monsieur le sénateur Didier Rambaud du groupe RDPI pour cinq minutes chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, ce n'est pas si souvent que nous arrivons au bout d'une discussion budgétaire au Sénat, qui plus est lorsque le nombre d'amendements déposés, 1740 1741 dépasse tous les records et six heures mes chers collègues, que tous les groupes et et pris leurs responsabilités jusqu'en début d'après-midi pour respecter le délai de l'ordre du jour, ce projet de loi de finances pour 2023 contient des choses positives pour les ménages, comme pour les entreprises, mais en cette semaine du congrès de mer je pense d'abord aux collectivités que nous devons soutenir, accompagner le gouvernement il y a, il est attentif puisqu'il décide d'augmenter en 2023 la dotation globale de fonctionnement de 320 millions d'euros après des années de baisse, et le maire et président d'interco que j'ai été entre 2001 et et 2017 s'en souvient, douloureusement, après des années de stabilisation entre 2017 et 2022 la DGF augmente pour la première fois depuis 13 ans une augmentation historique qui, soit dit en passant ne nous exonère pas pour autant de réfléchir à une réforme globale de la DGF pour ce pour que ces critères soient enfin plus lisible surtout plus compréhensible par les élus locaux, arrêtons-nous un instant aussi sur un autre point que contient ce projet de loi de finances ou plutôt cantonnée bien entendu je parle de la CVAE dans la réforme de suppression a été supprimé à la suite d'une situation ubuesque, chers collègues de la majorité sénatoriale, il y a dans votre position de l'incohérence, vous sortez de votre chapeau une idée de dégrèvement improvisé pour justifier votre report d'un an entre les réunions de commission et l'examen du texte en séance, résultats de des courses, on ne comprend plus, votre position sur le sujet, mieux encore, après avoir rejeté les amendements de suppression de la réforme de la CVAE, vous avez fait adopter votre report d'un an votre dégrèvement pour ensuite rejeté l'article que vous aviez pourtant modifié : où est la cohérence dans ses votes ne souhaitez-vous plus baisser là les impôts de production pour améliorer la compétitivité de nos entreprises, cette suppression devait pourtant profiter à 530000 entreprises dont 25 % des gains se réfléchis vers l'industrie au pied du mur plus de majorité dans l'hémicycle, assumez vos positions ne les modules est pas à l'eau, j'espère de prochaines sénatoriales à propos de cohérence revenant également sur le filet de sécurité, monsieur le rapporteur général lors du PDSR 2022, vous affirmez que les critères d'épargne brute et de potentiel financier vous convenez vous avez rejeté tous les amendements qui proposait pourtant d'assouplir les seuils et je vous cite : quand vous refusiez nos amendements au PLFR dernier si des communes échappent aux dispositifs, c'est que leur situation n'est pas aussi difficile que d'autres mais pour 2023 en plein congrès vous indiquer tout le contraire, affichant votre détermination à lever tous les critères les critères du filet sont perfectibles, il est impératif de l'assouplir, c'est ce qu'a déclaré, d'ailleurs tout à l'heure au congrès des maires, la première ministre et nous sommes heureux qu'un consensus puisse se dégager à ce sujet, mais il reste impératif de cibler le soutien sur les collectivités les plus fragilisés, nous espérons pouvoir y revenir en nouvelle lecture, à moins que le Sénat ne fasse un énième refus d'obstacle avec la l'adoption d'une question préalable qui tient désormais plus de la mauvaise habitude que d'un véritable positionnement politique de fond car ce dispositif, nous avons souhaité l'améliorer et complété par l'amortisseur sur les prix de l'électricité qui permet de réduire la facture de 20 % nous voulons qu'contribue à préserver les finances des collectivités, j'ajoute qu'en réalité nous réglerons ces difficultés lorsqu'on lui au niveau européen, nous arriverons à décorer le prix de l'électricité du prix du gaz et surtout lorsque notre pays sera souverain d'un point sur le sur le plan énergétique aujourd'hui dans l'urgence, notre groupe considère que l'État doit soutenir les collectivités les plus impactés notre groupe considère que l'État est au rendez-vous si l'on prend en compte l'ensemble des dispositifs, mes chers collègues, compte tenu des amendements adoptés sur la CVAE sur l'indexation de la DGF et son fils et son filet de sécurité, notre groupe RDPI s'abstiendra sur cette première partie du projet de loi de finances 2020 pour 2023 je vous remercie. Merci, chers collègues, je vais mettre aux voix l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances pour 2023, au terme de l'article 59 du règlement, le scrutin public et de droit, il va être procédé à son déroulement dans les conditions prévues par l'article 56 du règlement, le scrutin est ouvert.

Le scrutin est donc clos. Six voici le résultat du scrutin numéro 68, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs aux groupes politiques et notifié à la présidence Nombre de votants : Nombre de suffrages exprimés 307 pour l'adoption 216 contre 91, le Sénat a adopté président vénale, je vous demande d'intervenir à ce stade. Oui merci madame la présidente, mes chers collègues, donc en raison du retard pris lors de l'examen, donc de la première partie du projet de loi de finances et conformément aux règles de discussion budgétaire adopté par la conférence des présidents du Sénat, nous pourrions un accord avec le gouvernement, procéder aux modifications de lors de d'examen d'émissions suivantes : l'examen des missions, plan de relance et investir pour la France de 2030 serait reportée en dernier point de l'ordre du jour du vendredi 25 novembre l'examen des missions Engagements financiers de l'État et remboursements et dégrèvements serait lui reporté en dernier point de l'ordre du jour du mardi 29 novembre vous voyez que, malgré le retard pris, nous essayons de vous sauver le samedi, j'attends vos remerciements. Remerciements collectifs, monsieur le Président, je vous informe, cher collègue que je suspendrai la séance à 20 heures l'ordre du jour appelle l'examen des crédits de la mission transformation et fonction publique du compte spécial Gestion du Patrimoine immobilier de l'État, de la mission Gestion des finances publiques de la mission Crédits non répartis de la mission régimes sociaux et de retraite,

Mais la parole est à monsieur Claude nous un rapporteur spécial de la commission des finances. Pour cinq minutes. Bonsoir, monsieur le sénateur, Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues. Alors qu'il me revient de vous présenter des crédits de la mission Gestion des finances publiques, je ne peux commencer cette intervention sans rendre hommage au chef de brigades de vérification de la des défis du Pas-de-Calais tués dans l'exercice de ses missions, lundi, nous adressons avec Albéric de Montgolfier, co-rapporteur toutes nos pensées à sa famille et à ses collègues. En tant que rapporteurs spéciaux nous saluons chaque année dans notre rapport budgétaire le travail des agents du ministère de l'Économie et des Finances ces administrations ont démontré leur capacité d'adaptation et de transformation en menant d'importants projets à leur terme, cela ne veut pas dire, Monsieur le Ministre, coup, nous n'avons pas quelques points de divergence sur le budget qui nous est présenté, si nous avions l'habitude de dire que la mission Vincent des finances publiques était une des seules à contribuer à la rationalisation de la dépense publique ne pourront pas le faire cette année, les crédits atteindraient dit 10 6 milliards d'euros avec une hausse inédite, on n'en avait pas l'habitude de 5 IV, le contexte est donc clairement plus à la maîtrise des dépenses publiques, si même le ministère de l'Économie et des Finances dévie de sa trajectoire habituelle, seul point de satisfaction, le schéma d'emploi de la mission continue diminuer pour tenir compte de la numérisation et des gains de productivité suscitées par les réformes engagées ces dernières années, le rythme ralentit, certes, mais c'est après d'importants efforts en particulier de la part de la direction générale des finances publiques. Pour ce qui concerne les politiques menées par la DGFIP par la douane ou par le secrétariat général du ministère, le mot d'ordre semble être celui de poursuivre les chantiers entamés ces 5 dernières années années citerai un exemple avec le réseau de proximité de l'administration fiscale veut, c'est que c'est un point très important pour beaucoup d'entre nous, en particulier dans les territoires ruraux, il faut être clair : tous nos concitoyens ne sont pas en mesure de réaliser leurs démarches en ligne ou de pouvoir trouver la réponse est leur interrogation sur le site de la DGFIP, ils ont parfois besoin d'un point de contact de réponse particulière la numérisation ne doit pas conclure à l'exclusion, il en va de même pour le soutien apporté par les agents des finances publiques, aux élus locaux, à travers la mise en place des conseillers aux décideurs locaux, les retours sont globalement positifs mais encore faut-il que nombre suffisant d'entre eux soient déployés sur le territoire, il faut arriver à concilier présence dans les petites communes qui ne disposent souvent pas de l'expertise financière nécessaire et présence dans les grandes métropoles, avec les enjeux financiers les plus importants. Quelques mots désormais sur les 2 programmes de la mission Crédits non répartis le programme 551 provisions relatives aux rémunérations publiques a de nouveau fait l'objet cette année d'une ouverture de crédits à hauteur de 80 millions d'euros, le recours à cette dotation pour financer des mesures pourtant décidé plusieurs mois avant la programmation budgétaire semble devenir une habitude pour le gouvernement, or il est particulièrement regrettable du point de vue de la bonne information du Parlement que la ventilation des crédits demeure inconnue jusqu'à la fin des débats parlementaires, nous vous invitons donc le gouvernement à prendre au plus vite les mesures de répartition de ces crédits. J'en viens maintenant à dotation pour dépenses accidentelles et imprévisible qui fait l'objet cette année d'une ouverture de près de 1,8 milliards d'euros en CP, soit 14 fois le montant ouvert depuis 2018 ce montant nous paraît particulièrement déraisonnable au regard de l'exécution budgétaire des années 2021 et 2022, qui n'ont donné lieu à l'exécution d'aucun crédit sur cette dotation malgré le contexte économique et sanitaire incertain, c'est pourquoi nous avons déposé au nom de la commission des finances un amendement visant à minorer d'milliards d'euros, les crédits de ce programme, en tout état de cause, nous souhaiterions que le ministre-nous présentent davantage de justifications sur les raisons qui ont poussé le gouvernement à prévoir une dotation aussi démesuré que la crise énergétique et les incertitudes liées au contexte macro- économique internationale ne saurait selon nous justifier, pour conclure, il me revient de vous exposer la position de la Commission, ce ces de missions, nous vous proposons d'adopter les crédits de la mission Gestion des finances publiques, ainsi que ceux de la mission Crédits non répartis sous réserve bien sûr de l'adoption de l'amendement de la commission, je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur spécial j'appelle maintenant Monsieur Albéric de Montgolfier, rapporteur spécial de la commission des finances, et vous avez 5 minutes chers collègues. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, c'est de la commission des finances, mes chers collègues, avec Claude nous a, nous suivons également depuis plusieurs exercices, la mission transformation et fonction publique doté d'un milliard 100 millions d'euros notre constat est malheureusement le même chaque année, les projets portés par la mission sont nombreux mais la gestion, et souvent décevante la sous, consommation des crédits demeurent importantes sur certains programmes comme celui portant sur le fond de transformation de l'action publique et des il est dès lors très difficile d'apprécier la prévision des crédits pour l'année à venir quand on se rappelle les difficultés passées sur les contrats dans le cadre par exemple de la rénovation des cités administratives de l'État, les marchés ont mis plusieurs années être conclu résultat d'année en année, les délais de livraison sont repoussés. Autre conséquence, le coût des matériaux augmenter, obligeant ainsi l'État à procéder à des arbitrages, nous saluons toutefois avec Claude, nous, à la création de l'action résilience destinée à financer les gains action rapide, ce sont des actions à faible coût, qui génère de très importantes économies d'énergie, il s'agit pour nous d'une mesure d'une bien meilleure gestion que celle prévoyant par exemple, c'est de renforcer les effectifs de la Direction interministérielle de la fonction publique, on n'a pas très bien perçu l'intérêt d'une augmentation de ses effectifs, nous comprenons également encore mal son articulation avec des corps de conseils et de contrôle que les inspections générales il y en a suffisamment je pense pour ne pas avoir besoin de renforcer encore les effectifs, enfin, alors que la mission comprend bien l'intitulé Fonction publique : il est difficile d'identifier l'action du gouvernement à la en la matière, or bien sûr, réforme de la haute fonction publique sur les effectifs, cela a été dit longuement, notamment de la discussion générale en début d'examen de ce projet de loi de finances, rien n'est fait sur la rémunération, on reste sur des ajustements catégorielles ou des gré des arbitrages, j'en viens maintenant au crédit du compte d'affectation spéciale Gestion du Patrimoine immobilier de l'État, ces dépenses passerait de 416 millions à 340 millions d'euros 22 et 2023 ces diminutions concernent les opérations structurantes et les cessions tandis que les dépenses d'entretien du propriétaire augmente, elle devrait atteindre 200 millions d'euros en 2025 contre 155 millions aujourd'hui, pour une fois, c'est une source de d'intérêt de réjouissance puisque l'entretien l'entretien des bâtiments de l'État a longtemps été et reste le parent pauvre de la politique immobilière de l'État, les recettes du casse bête structurellement l'augmentation à hauteur de 490 millions d'euros en 2023 serait suivie d'une diminution à hauteur de 340 millions d'euros en 2024 et 2025 leur répartition est préoccupante en finançant aux 2 tiers les dépenses des produits par des dépenses pas des produits de cession, il y a évidemment une érosion progressive, une région excessive du Patrimoine immobilier d'État qui pourraient survenir et qui entraînerait les recettes du casse dans une spirale baissière. Si la politique de redynamisation des redevances domaniales était cet égard louable, on a peine encore en percevoir les fruits au-delà d'utilisation de ces crédits le casse-demeure contourner dans ces règles, tant par les dérogations à la mutualisation des produits que par le système d'avance sur cession du fait de l'insuffisance de ses recettes, le compte à midi d'affectation spéciale est également concurrencé par d'autres vecteurs budgétaire la mission transformation des fonctions publiques ou le plan de relance, je salue toutefois les initiatives lancées, que ce soit pour calculer le loyer des occupants ou pour valoriser les biens inoccupés, au total, si le cas ce n'est pas dans son état actuel suffisant pour porter les grands projets immobiliers de l'État, il n'est pas interdit d'envisager une réinvention de ce modèle, le chemin est étroit mais il existe, il faudrait sans doute inventé une véritable politique immobilière de l'État dans ce pays un État qui, encore une fois, utilise des méthodes un peu traditionnel, alors qu'il est d'un très gros propriétaires, pour conclure, il me revient de vous exposer la position de la Commission sur l'émission sur le casse-nouveau boson, compte tenu des modestes efforts d'adopter les crédits, la situation est loin d'être optimales mais je salue Monsieur le Ministre et je lui redis la situation est loin d'être optimales, mais nous devons conduire compte des progrès accomplis, donc c'est un encouragement que qu'un blanc-seing que nous vous êtes merci beaucoup. Merci madame Sylvie Vermeillet, rapporteur spécial de la commission des finances pour cinq minutes chers collègues. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la France se consacrent 13 6 % de son PIB au financement des retraites soit 3 345 milliards en 2021, c'est moins que l'Italie 15 6 % mais c'est plus que la plupart des pays de l'OCDE, dont l'Allemagne, la Belgique ou l'Espagne qui sont en dessous de 11 l'actuel équilibre de notre système de retraite devrait se dégrader dès 2023 jusqu'au milieu des années 2050, dans le meilleur des cas, si l'on s'accorde à éviter la baisse du niveau des pensions et la hausse des prélèvements alors la dégradation des comptes rend la réforme indispensable, celle-ci devrait se limiter à une dimension paramétrique en jouant principalement sur 2 critères pouvant être combinés une majoration de l'âge d'ouverture des droits de 62 à peut-être 65 ans, d'ici 2031 il y a une progression de 4 mois par an, l'accélération de la majoration de la durée de cotisation prévue par la réforme Touraine qui prévoit pour les personnes nées en 1973 ou après que la durée d'assurance requise pour l'obtention d'une retraite sans décote. Augmente progressivement d'un trimestre tous les 3 ans entre 2020 et 2035 pour atteindre 43 ans, soit 172 trimestres, mais il conviendra au préalable de s'entendre sur la convention d'équilibres choisi soit un effort de l'État constant en pourcentage de PIB, quel que soit le besoin du casse et des régimes spéciaux déficitaires, soit un équilibre permanent des régimes où l'État comble les besoins chaque année et c'est la convention actuellement retenus elle dicte un âge moyen de départ à 64 ans, dès 2030, portée à 66 5 ans d'ici 2000 60 pour atteindre le retour à l'équilibre du système. L'augmentation de l'âge de départ pose question au regard de la faible progression de l'espérance de vie, il en résulterait mécaniquement une moindre durée de retraite en effet les gains d'espérance de vie ne sont plus systématiques, une attention particulière doit aussi être porté à la pénibilité des métiers au dispositif carrières longues à la prévention de l'usure au travail, mais également à l'aptitude des entreprises à employer des seniors, le ministre de l'Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle, a indiqué que la réforme des retraites pourrait induire. 8 à 9 milliards d'économies au bout du quinquennat j'aimerais beaucoup disposer des éléments de calcul de cette estimation, je rappelle que la fermeture du régime des retraites de la SNCF a induit 4 virgule un milliards de mesures d'accompagnement donc de dépenses entre 2011 et 2020 et je me demande parfois pourquoi les syndicats redoutent tant ces réformes dans le détail la mission, la mission régimes sociaux et de retraite prend les régimes de retraite, des mines, de la à des régimes ferroviaires d'outre-mer de l'ORTF au programme 195 les régimes de retraite et de sécurité sociale des marins au programme 197 des régimes sociaux et de retraite des transports terrestres au programme 198 principalement ceux de la SNCF, de la RATP, mais aussi le réseau franco-éthiopien, qui compte 3 pensionner je déplore qu'il manque toujours dans ce périmètre, les régimes de l'Opéra de Paris, de la comédie française des industries électriques et gazières des non- salariés agricoles, des avocats et clair et employé de notaire en tout 5 4 milliards de contributions qui échappe à la mission, cela nuit considérablement à la lisibilité du système et par conséquent à celle d'une prochaine réforme la dotation 2023 de l'État envers les régimes de la mission devrait s'élever à 6 14 milliards en AP et en CP, dont 3 5 milliards pour la SNCF et 0,8 milliards pour la RATP, mais selon moi, ces prévisions sous-estime l'impact de l'inflation, par ailleurs, le compte d'affectation spéciale Pensions retrace les opérations relatives aux pensions civiles et militaires de retraite et d'invalidité des agents de l'État, les dépenses sont estimés pour 2023 à 64,36 milliards d'euros en AP et en CP. Dont 94 % pour les seules pensions civiles et militaires, en progression de 5,33 par rapport à la et les filles 2022, elles intègrent les évolutions du 1er juillet dernier avec la majoration du point d'indice de la fonction publique qui permet de doper les cotisations, mais pas autant que le coût de revalorisation des pensions, le PLF 2023 prévoit un solde négatif du CAS pension de 789 4 millions la baisse des effectifs cotisants elle niveau croissant des pensions ne peuvent que renforcer. Le déficit du CAF du casse, j'attire votre attention sur le fait que les taux de contribution employeur qui assure historiquement l'équilibre du CAS ont toujours permis de dégager des soldes excédentaire. Ces taux n'ont pas été révisée depuis 2014 et pour la première fois l'exercice 2022 devrait se clôturer par un déficit de 224 millions d'euros ainsi sans révision avec la hausse du taux d'employeurs, le solde excédentaire cumulé sera consommé d'ici 2025 la réforme devra se pencher sur ce déséquilibre croissant avec ses observations, je vous propose d'adopter l'ensemble des crédits de la mission

la commission des affaires sociales, partage en grande partie la position qui a été adopté par Madame la rapporteure effectivement en ce qui concerne le casse-régimes sociaux qui porte sur 6 milliards avec de régimes qui sont particulièrement concernés, à savoir la SNCF et la RATP, la SNCF, c'est déjà un régime fermé, donc quand on parle de suppression du régime ben ma foi, il y a déjà un certain nombre de mesures qui pourraient être prises avant et notamment un rattrapage par rapport aux âges parce qu'on a des âges de départ en retraite qui mérite qu'on s'y penche rappeler que la participation de l'État est au-delà de 60 % en ce qui concerne ces 2 régimes, ce qui est tout à fait important, c'est la raison pour laquelle nous avons émis un avis favorable mais avec un certain nombre de réserves, en ce qui concerne le casse-pension, là c'est un peu plus élevé puisque 64 milliards d'euros, ça concerne les fonctionnaires de l'état aussi bien civiles que militaires et nous avons déjà alerté depuis nombre d'années, en accord avec la commission des finances sur la dégradation de de ses comptes, compte tenu notamment du vieillissement démographique, alors certes, il y a un excédent la de 10 milliards qu'a un excédent d'ailleurs comptable, hein, il y a pas 10 milliards dans la caisse, parce que le gouvernement serait déjà attachés à les ponctionner, comme il l'a fait dans d'autres domaines, on l'a bien vu à travers ce PLF mais il n'empêche que ces 10 milliards vont s'évaporer au fil du temps puisque, dès 2025 le compte va être déficitaire, donc plus que jamais, il est important de prendre des mesures Monsieur le Ministre, c'est la raison pour laquelle, si on a mis un avis favorable, a avec un certain nombre d'inquiétudes, rappeler que les participations de l'État sont importantes, 74 % en ce qui concerne les civils 126 % en ce qui concerne les militaires et dans le cas d'un régime par répartition, il est plus que jamais important de l'parce que si c'est la dette qui paye cela hé bien c'est une mise en cause même du régime par répartition et Monsieur le Ministre, vous nous avez reproché de n'être 4 milliards sur les deux des entreprises tout à l'heure, et là on vous reprocherait de mettre des dizaines de milliards sur le dos de nos enfants demain, si on ne prend pas les mesures nécessaires pour équilibrer le système de retraite, le Sénat a pris ses responsabilités au gouvernement de les prendre maintenant, je vous remercie. Merci enfin Madame Catherine Di Folco, rapporteur pour avis de la commission des lois. 3 minutes chers collègues. Madame la présidente, messieurs les Ministres, chers collègues, l'année 2022 a été marquée par d'importantes mesures de revalorisation salariale dans les 3 versions de la fonction publique en résulte notamment une forte hausse de la masse salariale de l'État, qui atteindra 143 milliards d'euros en 2023, soit une augmentation de 5,35 % par rapport à 2022 rappelons également que, à rebours de l'engagement pris lors du quinquennat précédent le gouvernement vise désormais la stabilité des effectifs de la fonction publique de l'État comme vous le savez le programme 148 Fonction publique finance ses actions interministérielles, en matière de formation d'action sociale et de gestion des ressources humaines, il s'établit à 200 295 52 millions d'euros en autorisations d'engagement dans le PLF 2023 contre 303 25 millions d'euros en loi de finances initiale 2022 cette baisse apparente des crédits s'explique par la suppression du fonds d'accompagnement interministériel aux ressources humaines, créé en 2019, qui n'a pas fait la preuve de son efficacité depuis s'agissant de formation, je salue l'effort pour développer les classes préparatoires talent du service public qui ont remplacé en 2021, les classes préparatoires intégrées à la rentrée 2022, on compte 100 classes de ce type, qui accueille 1953 élèves par ailleurs l'expérimentation des concours Talents se poursuit en vue de son évaluation au 1er semestre 2024 en ce qui concerne l'action sociale interministérielle est prévue pour 2023, l'augmentation du montant des prestations individuelles et collectives, en raison de l'accroissement du nombre de bénéficiaires, je regrette que les indicateurs de performance relatifs à l'action sociale interministérielle et été remplacé depuis l'an dernier par un indicateur unique relatifs au taux de satisfaction des bénéficiaires, cet indicateur très subjectif, me paraît nettement moins pertinent, afin de permettre une évaluation précise des dispositifs d'action sociale interministérielle je vous proposerai donc un amendement visant à rétablir les 2 indicateurs de performance qui existait auparavant, enfin à l'heure où la question de l'attractivité de la fonction publique se pose avec une acuité particulière : la politique de ressources humaines des employeurs publics devraient constituer un levier majeur d'amélioration, or les actions prévues pour 2023, par exemple, pour améliorer la visibilité de l'emploi public semble encore timide, je suis pourtant convaincu qu'il y aurait un moyen efficace d'attirer davantage de candidats, et notamment des jeunes vers la fonction publique à travers le développement de l'apprentissage, à ce titre, je salue l'engagement pris par le gouvernement de poursuivre en 2023, le soutien de l'État à hauteur de 15 millions d'euros en faveur de l'apprentissage dans la fonction publique territoriale, en revanche, l'introduction dans le PLF de l'Arctique 40 sex IS rendant la participation de l'État et celle de France compétentes France compétences facultatives, n'est pas acceptable et nous en reparlerons Monsieur le Ministre, dans quelques jours, lors de l'examen des articles non rattachés sans ce soutien, l'équilibre du nouveau système de financement de l'apprentissage dans la fonction publique territoriale ne pourra être garantie sur le long terme, sous réserve de l'adoption de l'amendement évoqué la commission des lois a émis un avis favorable aux crédits du programme 100 qui vous remercie. Je vous remercie madame la rapporteure dans la suite de notre discussion, je vous rappelle que le temps de parole attribués à chaque groupe pour chaque unité discussions qu'on prend le temps d'intervention général et celui de l'explication de vote par ailleurs le gouvernement dispose au total de 10 minutes pour intervenir, la parole est à monsieur Éric Bocquet, du groupe communiste pour 4 minutes chers collègues. La présidente, messieurs les Ministres, chers collègues, cette année, nous avons le droit, dans le cadre de la mission Gestion des finances publiques a de rapports qui nous parviennent de l'Assemblée nationale, un 1er du rapporteur spécial monsieur Louis Margueritte, ancien directeur de cabinet de Monsieur, directeur adjoint du cabinet de Bruno Lemaire et de l'autre, celui de la députée Charlotte Leduc, tous 2 se sont penchés sur cette question cruciale : quels moyens sont consacrés au recouvrement de l'impôt, autrement dit à s'assurer que ceux qui sont redevables d'un impôt la quitte effectivement comment ne pas se réjouir d'une augmentation des crédits de 5,42 pour 100 en moyenne pour chacun des programmes que compte la mission parce qu'à bien y regarder, le programme 218 conduite et pilotage et politique, économique et financière porte une hausse des crédits de 80 millions d'euros, c'est une gauche de PME, des crédits de paiement servira pour 50 millions d'euros à la prestation d'appui et de support des cabinets de conseil viendront s'occuper de la sécurité juridique des services d'impôts, ce sont non moins de 210 millions d'euros engagés pour ces missions soient plus 61 % pour 2022, de l'autre côté, dans son rapport de mission Madame Leduc, constate, je cite une baisse alarmante des effectifs et la mise en place mal avisé des nouvelles technologies. Ne soyons pas trop dur 7 équivalents temps plein sont pourtant prévue dans le domaine du conseil en stratégie depuis 2018, c'est plus de 1000 emplois qui ont été supprimés au service du contrôle fiscal, précisément, selon la DGFIP, grâce au recours à l'Intelligence artificielle pour le ciblage de la fraude et la valorisation des enquêtes, des gains de productivité, voilà l'objectif central de notre gouvernement, pourtant, nous ne cesserons de le répéter : les robots ne remplaceront jamais les humains, ils les aident et les assistent, dans le meilleur des cas, cette trajectoire est critiquable et conduit à l'échec de la mission à l'abaissement du plafond d'emplois de 863 équivalents temps plein travaillés, les transferts de mission de la Direction des douanes au profit de la DGFIP exigerait des recrutements, en conséquence nous nous félicitons du ralentissement du calendrier et de la redéfinition des missions transférées, c'est sans doute grâce aux mouvements sociaux dans les services de la douane qui a été enrayer cette machine infernale qui nie les compétences des uns et des autres et invisibiliser les spécificités de recouvrement, l'expertise propre au métier des agents comme pour pallier ces carences en personnel, le rapporteur spécial de la majorité présidentielle appelle, je cite, à conforter la relation de confiance entre la DGFIP et les entreprises qui permet à la fois de sécuriser le recouvrement des prélèvements obligatoires, derrière cette nouvelle idéologie se cache le nouveau mantra de la Start-Up fiscal la technologie et cette nouvelle doctrine ainsi que les baisses d'effectifs et l'inflation des dossiers explique probablement la chute des droits et pénalités notifié par rapport à 2012 de moins 4 2 milliards d'euros et des sommes encaissées relativement stable, le juge Van Ruymbeck, le sait mieux que quiconque les fraudeurs, dit-il, ont toujours un coup d'avance, mais il pense comme moi et d'autres ici que l'évasion fiscale n'est pas une fatalité, je vais citer, je pense que le jour où on s'attaquera vraiment au paradis fiscaux aux outils, aux sociétés Offshore, on mettra au pas ces paradis fiscaux, ce message d'espoir, doit être entendu, il doit nous permettre d'opérer un virage dans la doctrine, les moyens et des règles politiques fixé à l'endroit de ceux qui se détournent de l'impôt et de ce qui rentre ce phénomène possible, c'est un impératif pour qu'il devienne impossible de prononcer la main sur le coeur pour une multinationale qui fuient l'impôt, nous sommes fiers de nous conformer aux règles fiscales des pays où nous opérons, je vous la ferai pas en anglais, le français est la langue de la République, merci. Merci, cher collègue, la parole est à présent à monsieur Michel Canet va être pour l'Union centriste 4 minutes lutte chers sénateurs. Merci madame la présidente, messieurs les Ministres, chers collègues, je remplace au pied levé notre collègue Vincent Delahaye, qui aurait bien voulu vous délivrer aujourd'hui un certain nombre de messages, je vais tâcher de le faire à sa place, tout d'abord je voudrais souligner le propos tout à l'heure de rapporteur spécial, Sylvie Vermeillet, qui a évoqué les régimes spéciaux, va sans doute pas s'étendre là-dessus mais vous rappeler que, aujourd'hui, il y a quand même des régimes spéciaux de la SNCF et de la RATP qui mobilise 4 milliards de fonds publics, si l'on met ça en rapport d'un milliard et demi qui sont mobilisés pour le filet de sécurité, énergie, vous imaginez le l'impact budgétaire concernant la fraude fiscale, si on peut se réjouir, effectivement, qu'il y a des progrès qui a été réalisé dans la lutte contre cette fraude fiscale, il reste encore, et notre collègue Nathalie Goulet est là pour, je dirais, de donner un certain nombre de pistes de travail, il reste encore beaucoup à faire au niveau de la fraude sociale et on espère qu'effectivement le gouvernement soit particulièrement attentif à tout cela, alors si l'on devait juger le niveau du bonheur à l'importance de la dépense publique qui était fort en en France, on peut se référer au rapport que publie les Nations unies à cet égard, et il est instructif puisque, on constate que de nombreux pays, comme la Suisse, l'Islande ou encore les Pays-Bas enregistrent un score de bonheur supérieur à la moyenne des pays de l'OCDE, avec un secteur public de taille inférieure à la moyenne et la France, quant à elle avec un secteur public de taille très supérieur à la moyenne, hélas, est largement en dessous de la moyenne, donc il faut que nous soyons modestes sur le sujet et que nous pensions à ce que le bonheur ne se résume pas à l'importance des moyens budgétaires que l'on dédie à l'action publique alors sur cette mission je salue le les rapporteurs, Claude Mougin et Albéric de Montgolfier pour ce qui concerne le Patrimoine immobilier ou de ressources humaines, nous n'avons pas tout à fait c'est faut le dire la la même conception de de la gestion,

rendu aux citoyens, il faut que l'on continue là-dessus notamment à ça en faisant en sorte que cette numérisation permet d'économiser sur les moyens de fonctionnement, en particulier en personnel pour optimiser nos dépenses la dépense publique, elle, elle reste encore extrêmement forte, il faut le dire et le regretté sur les questions de des effectifs de la fonction publique, parce que quand on constate que la population depuis 81 a augmenté de 18 % dans notre pays pendant ce temps là, les effectifs de la fonction publique ont augmenté de 40 40 % c'est dire les évolutions contrastées des choses, monsieur le Ministre de la fonction publique et là aussi le groupe de l'Union centriste appelle à ce que nous soyons le plus vigilants possible pour éviter que ces dépenses de personnel ne grève effectivement de dépenses publiques, parce que ce sont des dépenses récurrentes et on voit bien qu'on a la difficulté à l'équilibre de nos comptes, dans ces conditions, avec des dépenses de personnel qui sont particulièrement élevés, et en particulier, on note que dans notre pays, les contrats à durée déterminée ou les je dirais en statut de de, on ne voit pas de la ascenseur publics sont de 20 % en France contre 60 % en Allemagne contre 85 % en Italie 92 % au Royaume-Uni 99 % en Suède, peut-être que nous aurions beaucoup plus de souplesse à revoir ce statut de la fonction publique pour, je dirais, ne pas systématiquement titularisé, tout le monde, voilà donc quelques observations que je souhaitais faire en tête du groupe de l'Union centriste, vous remercions de votre attention. Merci, la parole est à présent à monsieur Stéphane Artano pour le groupe RDSE pour 4 minutes chers. Madame la présidente, messieurs les Ministres, Monsieur le président de la commission des finances, mesdames, messieurs les rapporteurs, chers collègues, je n'ai que quelques minutes pour évoquer les enjeux de 4 émissions et de de comptes spéciaux étant dans l'incapacité de les traiter dans ce délai j'apporterai principalement des observations sur l'émission afin d'éviter les répétitions sur le chiffre qui serait pas forcément toujours très intéressant, je commencerai par la mission Gestion des finances publiques, qu'on vient de saluer d'abord l'augmentation des crédits qui c'est dans la mission s'élève à 10 milliards 5, soit une hausse de plus de 5,4 % cette hausse est donc la bienvenue dans un contexte où les administrations financières sont au coeur d'importantes transformations en effet le renforcement des moyens de lutte contre la fraude fiscale doit être une priorité au regard des marges de progrès existantes, toutefois, il faut rester attentif aux objectifs qui seront définies dans le comme de la DGFIP à venir pour la période 2023 2027 on parallèle, la poursuite du développement des outils de Data Mining et d'Intelligence artificielle, doit aussi permettre de renforcer les capacités d'analyse des administrations face à la complexification de la fraude de plus il est nécessaire de compléter l'effort d'information des parlementaires en renseignant les effets des réformes conduites au sein des administrations financières sur les emplois, en particulier à la DGFIP, j'en viens maintenant à la mission Crédits non répartis où je note que la provision relative aux rémunérations publiques, j'ai de nouveau l'objet d'une ouverture de crédits à hauteur de 80 millions d'euros destinés à financer l'extension du forfait mobilité durable ce qui est une bonne chose, par ailleurs, au même titre que l'amitié, la commission des finances, j'aurais quelques retenues sur l'augmentation excessive des crédits de la dotation pour dépenses accidentelles ou imprévisible, c'est le vont tout de même à près de 1,8 milliards d'euros ne gouvernement justifie cette hausse. D'une enveloppe 14 fois supérieure au montant qu'on de 124 millions d'euros sur les seules incertitudes liées à la crise énergétique et au contexte international et macroéconomiques, dont acte, je poursuis avec le budget de la mission transformation et fonction publique qui se décompose, est désormais en 6 programmes n'a vocation interministérielle qui concernent des sujets aussi variés que la rénovation des cités administratives de l'État, des projets porteurs d'économie à moyen terme, les ressources humaines ou encore les Start-Up d'État je souhaite porter l'accent sur les crédits proposés pour le programme Fonction publique qui s'établit à hauteur de 285 millions d'euros, ce montant traduit une légère baisse par rapport au budget de l'année dernière mais se maintient tout de même à un niveau élevé lorsqu'on s'intéresse à l'évolution pluri-annuel, quelques mots sur le remplacement de l'ENA et de par l'INRP si dans l'ensemble, cette réforme paraît aller dans le bon sens dans ces grands objectifs plusieurs points d'intentions doivent néanmoins être souligné, il convient donc d'être essentiel et de veiller au maintien d'un haut niveau de professionnalisation du corps préfectoral, de plus il ne faut pas oublier que la mise en extinction du corps diplomatique a été mal vécue par qui et d'Orsay, ce qui risque d'affecter la qualité et le rayonnement de notre réseau diplomatique, il est important d'y apporter des garanties, enfin, comme l'a révélé la récente commission d'enquête du Sénat les recours au cabinet conseil par l'État, soulève des questions fondamentales qui intéressent directement la fonction publique, la tendance croissante à externaliser en dehors de l'administration, la réflexion portant sur les politiques publiques, interroge la capacité de notre État à disposer des compétences nécessaires à la réalisation de ses missions les plus essentiels, en effet, le recours au cabinet conseil doit être mieux encadré, rendu plus transparent et il paraît important de prévoir dans la loi que ces cabinets soit soumis à des obligations déontologiques ne reviendrait pas sur les comptes spéciaux qui ont déjà été largement abordé en conclusion de messieurs les Ministres Monsieur secrétaire : le groupe RDSE votera les crédits de ces 4 missions et de ce de comptes spéciaux contenus, l'importance des enjeux qu'il soulève. j'appelle à présent monsieur Cyrille pelle va pour intervenir au nom des républicains pour cinq minutes. Madame la présidente, messieurs les Ministres, Monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, nous débutons l'examen de la seconde partie du budget pour 2023 je m'arrêterai d'abord sur la mission transformation et fonction publique hein, pour laquelle je souscris aux conclusions des rapporteurs si la programmation est ambitieux, hein, ces dernières années l'exécution à peu suivi et d'importants retards ont été constatés sur le décaissement des crédits, à ce titre, je me réjouis qu'une nouvelle action résilience étaient incluses dans le programme 348 ans, dans le but de sélectionner des projets de rénovation à gain rapide, cela devrait permettre un décaissement accélérer, même s'il est permis de douter qu'il soit totale d'ici fin 2023 la problématique est la même pour le programme 349 ans avec le Fonds FTA dont l'évaluation de l'efficacité serait la bienvenue pour le programme Fonction publique : s'il faut se réjouir de la stabilité des crédits, je souhaite comme notre rapporteur pour avis alerter sur le défi, capitale de l'attractivité de la fonction publique, chacun d'entre nous a pu constater les difficultés de recrutement liées à ce manque d'attractivité par nos échanges sur le terrain, faute de réponse ambitieuse et rapide, hein, la pérennité de la fonction publique pourrait être compromise et avec elle la qualité des services publics, je tiens à rappeler que tous les territoires, ne sont pas logés à la même enseigne en face à ce défi et que des mesures différenciées visant à fidéliser les fonctionnaires et attirer de nouveaux talents de monter de prise en fonction des particularités des territoires, à ce titre, je proposerai des amendements visant à donner accès aux fonctionnaires de la Haute-Savoie à la prime de résidence de laquelle ils sont injustement exclu, alors que le coût de la vie et dans de nombreuses communes savoyardes, aussi, si ce n'est plus élevé que dans des villes d'autres départements ayant ayant je sais qu'il s'agit d'un sujet très spécifique, un local à ma circonscription, mais j'essaye, hein messieurs les Ministres, que vous saisirez cette problématique après des années d'alerte parlementaires du département à ce sujet, je m'arrête rapidement sur le compte d'affectation spéciale Gestion du Patrimoine immobilier de l'État, celui-ci enregistre une baisse de 18,2 % de ses dépenses, mais les dépenses d'entretien augmentent de 9,3 % nous pouvons nous en réjouir, mais à condition que l'exécution des crédits et bien lieu si les recettes sont exceptionnellement en hausse cette année, elles connaissent en réalité une baisse tendancielle et sont dus à une majorité à des cessions, ce qui pourrait conduire à une érosion du Patrimoine de l'État, à cet égard la politique de redynamisation des redevances et le recours aux baux emphytéotiques sont bienvenus, mais doivent monter en puissance, de toute évidence, le rôle d'impulsion stratégique du CRS n'est pas pleinement rempli est concurrencée par d'autres vecteurs budgétaires, ce qui entraîne un éclatement néfastes des objectifs des pistes devront donc être exposé pour y remédier, quelques rapides remarque également pour la mission Crédits non répartis son programme 551 n'appelle pas de commentaire particulier, si ce n'est qu'une répartition rapide des crédits vers les différentes missions et souhaitable et qu'il convient de mieux respecter le principe de spécialité budgétaire à l'avenir pour le 552 relatifs aux dépenses accidentelles imprévisible si les craintes du gouvernement sont justifiées, en ce qui concerne la crise énergétique et le contexte hein international et macro-économique, hein, il est évident que les crédits qui s'élève à plus de 1,7 milliards d'euros sont bien trop excessif, je souscris à ce titre à la proposition des rapporteurs visant à réduire d'un milliard, son montant en concernant la mission Gestion des finances publiques, j'ai bien pris note du fait que la hausse des crédits sur exceptionnelle et qu'elle vise à poursuivre les réformes engagées pour rationaliser des finances publiques, on s'appuyant sur l'informatique pour gagner en productivité et améliorer les contrôles fiscaux, objectif auquel je souscris, de même la réorganisation territoriale de la DGFIP est apprécié en ce qu'qui vise à augmenter ces points de contact mobile sa présence dans les villes moyennes et à continuer le déploiement du réseau, conseiller aux décideurs locaux, nous resterons cependant vigilants à ce que la répartition des conseillers soit équilibré pour finir avec la mission régimes sociaux et de retraite, ainsi que les 16 pension la dégradation des comptes ça doit conduire à augmenter l'âge de départ à la retraite, seule façon de les rééquilibrer mais le montant des économies attendues reste insuffisamment documenté ne garantissant pas la sincérité de la prévision budgétaire, en outre, l'optimisation des coûts de gestion et nécessaire pour pallier l'augmentation des dépenses de certains régimes en ce qui concerne plus spécifiquement le CSA, la progression des crédits et l'insuffisance des recettes doivent conduire à activer de nouveaux leviers en particulier l'évolution du taux de contribution employeur il pourrait notamment être pourtant de changer de méthode, en prévoyant un taux de cotisations patronales, doublée d'une subvention d'équilibre, de même la pertinence de la notion de technique devrait être étudiée et la création de véritables réserves affecté au F. R. R serait opportune, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à présent président Claude Malhuret pour le groupe des Indépendants et vous avez quatre minutes cher président. Madame la présidente, messieurs les Ministres, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, il est en France un paradoxe qui a la vie dure, les citoyens veulent à la fois plus de service public et moins de pression fiscale plus d'État et moins d'impôts, plus de dépenses et moins de recettes. Pour dépasser ce paradoxe, il n'y a guère qu'une façon d'avancer, c'est de réformer l'État, c'est une tâche de Sysiphe un travail continu auquel nous ne devons jamais renoncer réduire notre déficit tout en améliorant en ma qualité de nos services publics tels et donc notre mission, elle n'est pas impossible, le gouvernement l'a d'ailleurs prouvé notamment par le biais d'une réforme technique mais populaire, je pense à la mise en oeuvre du prélèvement à la source, les cases qui a coché toutes les cases, premièrement, elle a améliorer la qualité du service public rendu aux contribuables en simplifiant leur démarches deuxièmement elle a permis d'augmenter les recettes de l'État en actualisant les prélèvements par rapport aux revenus, troisièmement, il fait preuve d'efficience et mobilise moins de fonctionnaires à Bercy pour le suivi de ces procédures. Ainsi, transformer l'action permet à la fois d'améliorer les recettes sans augmenter l'impôt et de baisser les dépenses, sans dégrader les services publics, Monsieur le Ministre, messieurs les ministres, il faut bien l'avouer, nous aimerions tous ceux que cet exemple, puisse être suivi par l'ensemble de nos administrations, alors que le schéma global de la mission Gestion des finances publiques baissera sur l'année 2023 la qualité du service rendu doit rester au rendez-vous et les actions ont continué de se moderniser. C'est avec le même esprit de réforme que je souhaite aborder l'autre aspect de cette discussion qui concerne le compte d'affectation spéciale Pensions. Depuis que la réforme des retraites a été balayée par la pandémie, nous examinons chaque année ces crédits dans la crainte ou l'espoir, c'est selon, de son retour, désormais, la donne a changé et l'élection présidentielle, a confirmé que les Français sont prêts à une réforme du système de retraite, les contours de cette réforme, nous le verrons les contours de cette réforme reste à définir, le gouvernement a d'ores et déjà engagé une concertation avec les partenaires sociaux sur le sujet, il faudra désormais aller au bout et le plus tôt sera le mieux, le rapport spécial de notre collègue Sylvie Vermeillet nous le rappelle un recul de l'âge de départ à la retraite permettrait d'économiser entre 8 et 9 milliards d'euros au bout du quinquennat il faut bien sûr se défier des solutions miracle, le rapport du conseil d'orientation des recettes précise que le rehaussement de l'âge légal de départ en retraite peut également entraîner des dépenses supplémentaires pour l'assurance maladie, c'est pourquoi notre groupe prône une réforme globale plutôt qu'un ajustement paramétrique sur le seul levier de l'âge de départ, cette réforme devra également rouvrir le débat des régimes spéciaux, l'analyse de la mission régimes sociaux et de retraite, nous rappelle que le financement des de régimes spéciaux de la RATP, de la SNCF représente plus de 4 milliards d'euros ses crédits augmenteront de 5 % sur l'année 2023 enfin le compte d'affectation spéciale comme la mission régimes sociaux et de retraite ne constitue qu'une part des financements de l'État vers les régimes de retraite, au total, les dépenses publiques consacrées aux retraites représentent près d'un quart du total des dépenses publiques, soit 14 % du PIB. En attendant que ce débat n'arrive au Sénat, notre groupe votera en faveur des crédits, les différentes missions que nous examinons aujourd'hui. Merci, cher collègue, la parole est à présent monsieur Daniel Breuiller du groupe écologiste pour 4 minutes

notre groupe souhaite comme les rapporteurs exprimer tout d'abord son total soutien à la famille du chef de brigade décédé cette semaine dans l'exercice de ses fonctions, nous voulons également rendre hommage à sa collègue blessé et plus largement à tous les agents de la DGFIP à propos de la situation du contrôle fiscal, nous avons déposé un amendement 209 pour renforcer les moyens de ce contrôle fiscal en effet le nombre d'agents affectés dans les différents services de contrôle de la DGFIP a baissé d'un tiers, ces 10 dernières années de 13336 postes en 2010 environ 9000 9 % des effectifs de la DGFIP en 2020 dans le même temps, les résultats du contrôle fiscal se sont effondrés, le Fisc a notifié 21,2 milliards d'euros de redressements fiscaux en 2015 et 10 minutes milliards 10 7 milliards en 2021, cela représente une baisse de moitié sans doute en partie seulement expliqué par un système plus robuste, si la hausse des moyens informatiques fortement et soutient un choix stratégique une sans doute nécessaire, l'affaiblissement des moyens RH et constaté. Vous choisissez au nom de la modernisation de l'action publique, que ce ne soit plus par exemple les agents comptables des trésoreries de proximité qui encaisse les espèces de régie des communes, permettez moi puisque j'étais voilà encore si peu élu local de constater que aller à la Banque Postale signifie pour certaines collectivités de voir souscrire un contrat, un contrat privé de transport de fonds pour la sécurité des agents régisseur quand vous choisissez que des usagers aillent régler leurs factures, titré au bureau de tabac, vous affaiblissez à notre sens, le modèle du service public que nous souhaitons bien sûr, il y a la dématérialisation des paiements, c'est un choc de simplification bienvenue pour la plupart des familles, mais je veux vous le dire, il reste dans ma ville, encore 3 à 4 % de familles qui viennent régler leurs factures de cantine en mairie avec des pièces et ce n'est pas de gaieté de coeur, c'est le reflet d'une réalité de précarité auquel nos agents publics doivent également faire face, votre démarche par ailleurs ne parle pas tout à fait ses fruits puisqu'on voit dans le volet ressources humaines de cette mission, qu'il y a désormais dans ce secteur comme dans beaucoup de secteurs de la fonction publique, une véritable crise Merci, la parole est maintenant à ma Monsieur Dominique Théophile du groupe RDPI pour 4 minutes chers collègues.

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, c'est donc avec l'examen simultanée de 4 émissions que nous abordons la seconde partie du projet de loi de finances 2 pour 2023, c'est cette année encore, une invitation à la concision invitation que je m'efforcerai d'quelques d'quelques mots simplement pour vous dire que nous nous associons bien sûr à l'hommage qui a été rendu à l'inspecteur des finances publiques, tué lundi dernier dans l'exercice de ses fonctions et que nous apportons notre profond soutien à sa famille, à ses proches et à ses collègues, aujourd'hui plus encore, alors que nous nous apprêtons à débattre du budget de la direction générale des finances publiques les deux premières missions Gestion des finances publiques et transformation et fonction publique retrace les crédits qui participent activement à la transformation de l'action publique, elles s'inscrivent en cela dans la dynamique initiée il y a 5 ans par le président de la République, la première qui porte le les crédits de la DGFIP et de la DG DDI verra son budget augmenter sensiblement en 2023 autour de 11 milliards d'euros, en raison principalement de l'augmentation des crédits informatique et immobilier : nous nous réjouissons du bon déroulement de la réforme qui vise à unifier au sein de la DGFIP, le recouvrement des taxes ainsi que des conséquences positives de la réforme de son réseau de proximité, soulignant également les efforts déployés par ces 2 directions valoriser les données en vue de lutter plus efficacement contre la fraude, soulignant aussi le renforcement de la présence de la DG DDI à la frontière numérique alors que se développe de manière exponentielle, le commerce en ligne dernier motif de réjouissance, les crédits alloués à Tracfin pour renforcer sa capacité à traiter un nombre croissant d'informations connaîtront une forte hausse en 2023 la mission transformation et fonction publique aux traces, quant à elle, les crédits interministériels destinés à soutenir directement à la transformation publique elle connaîtra en 2023 une une montée en charge importante puisque le budget de cette mission c'est devra à 800 millions d'euros en autorisations d'engagement et à milliards d'euros en crédits de paiement, soit une hausse respective de 79 et 44 la mobilisation d'une enveloppe destinée à réduire les dépendance aux énergies fossiles, des bâtiments de l'État et de ses opérateurs le ré-abondement du Fonds pour la transformation de l'action publique qui permettra de générer des économies pérennes et la volonté du gouvernement de placer l'inclusion et l'expérience des de l'usager au coeur de la conception des services publics numériques, soulignant également le développement de l'apprentissage dans la fonction publique et le lancement du volet du CNR qui lui est consacré, ainsi que des efforts déployés par le gouvernement pour réduire les dépenses de prestations de conseil et renforcer la capacité de conseil interne de ces administrations quelques mots enfin sur la mission Crédits non répartis qui fait une nouvelle fois l'objet d'une demande de crédit afin de financer l'extension du forfait mobilité durable et des mesures de convergence des régimes indemnitaires indiciaire résultant de la création du corps des administrateurs de l'État, les crédits de cette mission reste cependant principalement porté sur le programme 552 dépenses accidentelles et imprévisible, avec une enveloppe de près de 2 milliards d'euros enveloppe dont nous aurons l'occasion de parler dans quelques instants, la mission régimes sociaux et de retraite, enfin,

d'un relatif consensus au sein de notre assemblée, je vous remercie. Merci, la parole est à présent Madame Florence blattes comptable pour le groupe socialiste, pour six minutes chers collègues. Je suspendrai la séance après cette intervention. Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'examen conjoint des missions Gestion des finances publiques régimes sociaux et de retraite et transformation et fonction publique est un exercice impossibles dans le temps qui nous est alloué, je me concentrerai donc sur les enjeux qui concernent plus directement les quelque 5 6 millions d'agents publics qui dans nos écoles, nos hôpitaux, nos commissariats nos collectivités exerce dans des conditions parfois difficiles, la nécessaire mission de service public je veux profiter de l'examen de ce budget pour saluer l'ensemble des agents de nos différentes fonctions publiques pour leur professionnalisme, leur engagement au service de nos concitoyens, la fonction publique fait aujourd'hui face à une crise du recrutement qui se constate dans tous ses versants. Avec des conséquences très concrètes sous le service rendu aux usagers, service horaires réduits, diminution du temps de présence au guichet et recours accru à la dématérialisation qui éloigne des services publics les plus précaires, les personnes âgées et qui alimente la mécanique de non-recours aux droits le défi de l'accessibilité de nos services publics passe donc nécessairement par une amélioration de son attractivité pour assurer aux usagers un service de qualité et de proximité, il faut des femmes et des hommes qui veuille s'engager dans la fonction publique, la crise de recrutement n'est pas une crise de vocation pour le service public est, elle s'explique plutôt par une perte de sens et une dégradation des conditions de travail au sein de la fonction publique, nourrie par le développement de la contractualisation de l'externalisation, la crise du recrutement s'explique aussi par la faiblesse des rémunérations, j'observe que nous partageons ce constat Monsieur le Ministre, puisque vous avez récemment déclaré que le déficit d'attractivité de la fonction publique est liée à la problématique salariale, le Parlement a certes voté une revalorisation de 3,5 % du point d'indice, mais cette augmentation intervient après 10 années de gel du point d'indice, hormis 2016, 2017 et dans son contexte inflationniste exceptionnel. Certes, il s'agit de la plus forte augmentation générale du point d'indice depuis les 40 dernières années, mais il s'agit aussi et surtout de la plus forte hausse de l'inflation depuis les 40 dernières années, cette augmentation aussi importante qu'elle soit ne couvre ni l'inflation pour 2022, ni la perte de pouvoir d'achat accumulées depuis 2017 en l'absence de nouvelles mesures générales sur les salaires, vous affirmez que les mesures de compensation individuelle devrait permettre de maintenir le pouvoir d'achat de la fonction publique, mais les compensations individuelles comme la garantie individuelle de pouvoir d'achat sont des mécanismes qui ne sont plus adaptées et qui ne sont pas à la hauteur en terme d'attractivité si avec les compensations individuelles, les agents sur la grille ne perde pas de pouvoir d'achat pour les fonctionnaires qui passent le concours, il n'y a pas de compensation individuelle et par ailleurs la grille et de moins en moins attractif par rapport aux possibilités qu'auraient les mêmes personnels dans le privé par ailleurs à l'action sociale interministérielle qui vise à améliorer les conditions de vie des agents et de leur famille, peut être un levier d'amélioration du pouvoir d'achat des agents publics, plus directement au budget qui nous est présenté ces crédits sont attendus en légère hausse, plus 1 virgule 8 pour % mais il reste faible en volume et cette hausse est bien entendu imputer par l'inflation, je prendrai 2 exemples, tout d'abord, les crèches, le dispositif qui permet aux agents de bénéficier prioritairement de places en crèches implantées dans les aires géographiques adaptées à leurs besoins, elle reste trop modeste, le montant global trente 7 millions est à peine plus important que les crédits ouverts par le budget précédent 30 1 1000000 et la quasi-stabilité freine nécessairement le développement du parc, seuls 100 places en crèches ont été créées en 2022, 2022, et il n'est, a annoncé que 135 places supplémentaires pour 2023 enfin une autre problématique : le logement des fonctionnaires, les chiffres du PLF montre l'absence d'une grande politique sociale interministérielle en matière de logement alors que le logement représente un poids toujours plus lourd dans le budget des Français, et cela concerne en particulier les fonctionnaires en 2020, lors du débat budgétaire pour l'année suivante, j'ai souhaité attirer l'attention, par un amendement sur la nécessité de réviser l'ensemble du dispositif de l'indemnité de de résidence ce dispositif comme vous le savez, n'a pas été modifiés depuis 2001, il est aujourd'hui obsolète, les montants proposés sont ridiculement faible et son périmètre doit également être révisée certaines zone frontalière ne sont pas incluses, alors qu'elles subissent des loyers très très élevé, je pense en particulier au Pays de Gex dans mon département, mais également à la Haute-Savoie les difficultés pour les fonctionnaires, pour se loger sont vraiment immense votre prédécesseur et le gouvernement s'était engagé devant le Sénat à revoir ce dossier, considérant que les politiques sociales, d'aide à l'accès au logement, permettent à des agents d'avoir accès à un logement adapté pour un coût connu et encadrée et donc, en dépit des relances malheureusement nous n'avons rien vu venir, Monsieur le Ministre, d'ailleurs, devant la commission des lois de l'Assemblée nationale du 26 octobre vous avez reconnu qu'il y a là un vrai sujet et je vous demande vraiment avec insistance, c'est important important pour un certain nombre de territoires, de passer enfin aux actes, je vous remercie. Merci à la présidente, oui, c'est une demande au nom du gouvernement, monsieur le président de la commission, vous avez annoncé tout à l'heure pour le calendrier des prochaines missions une un examen demain en fin de de d'du jour de la mission, plan de relance et investir investir pour la France de 2030 et un examen mardi en fin d'du jour de la mission Engagements financiers de l'État et remboursements et dégrèvements et on souhaiterait demander si cela est possible, l'inversion de ces 2 missions entre eux donc demain et mardi. Monsieur Président en mettent vous d'accord. Oui, madame la présidente, avec l'accord des rapporteurs spéciaux en charge en particulier : accord pour l'inversion et donc nous l'annoncerons évidemment tout à l'heure. Si il en est ainsi décidé, je vais suspendre la séance le sera reprise à 21 heures 30 pour la suite de l'examen de ces missions et comptes spéciaux, la séance est donc suspendu bonne appétit chers collègues.